Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Il n'y a pas d'observation d'ailleurs ce serait difficile. Le procès verbal est adoptée sous les réserves d'usage. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant Renault à revaloriser le statut de secrétaire de mairie. Présenté par Madame Céline Brulin, Cécile Cukierman Michelle Gréaume Marie-Claude var alias Éliane Assassi et plusieurs de leurs collègues. Dans la discussion générale. La parole est à madame Céline Brulin, pour le groupe CRCE, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre Madame la rapporteure chers collègues nous sommes jeudi. Il est 10h 30. La secrétaire de mairie de cette petite commune du Pays de Caux est arrivé en mairie à Elle y en poste chaque fin de semaine. Le reste du temps elle est dans une autre commune à une trentaine de kilomètres de là. Impossible en effet pour les petites communes de recruter des agents à plein temps pour ses collègues. C'est parfois entre 3 voire 4 communes qu'il faut se partager ce n'est pas forcément déplaisant mais pour peu que ces communes se situent dans des communautés de communes différentes. Cela multiplie les problématiques les sujets à traiter les enjeux à prendre en compte. Notre secrétaire de mairie a décidé de consacrer du temps ce matin à examiner l'opération 5000 terrains de sport. L'équipe municipale à un projet de City stade et lui a demandé de rechercher les subventions dans la commune pourrait bénéficier les éléments ont été envoyés fin février mais entre le budget à finaliser les réunions sur le plan local d'urbanisme intercommunal a organisé les tâches du quotidien à accomplir. Elle n'a pas encore eu le temps de s'y pencher. Problème, les dossiers doivent être déposés avant le 31 mai et ça peut faire cours pour aboutir le projet et sollicité les différents devis auprès des entreprises locales. Il faudra qu'elle en parle au maire. Il est au travail et ne viendra en Amérique en fin d'après-midi elle restera jusqu'en début de soirée pour pouvoir travailler avec lui. Plusieurs habitants arrivent en mairie leur connexion internet ne fonctionne plus. L'un d'entre eux étant télétravail. Il est un peu en colère car il ne va pas pouvoir assurer ses missions déjà qu'ici la fibre. Ce n'est pas pour tout de suite il a bien essayé de joindre l'opérateur mais il est tombé sur un répondeur comme souvent maintenant, tapez 1 tapez 2 veuillez répéter votre message, nous n'avons pas compris. Rien à faire, il n'a pas pu joindre il n'a pu joindre personne qui puisse l'aider alors vers qui s'est-il tourner la mairie qui est le premier mais parfois aussi le dernier des services publics dans nos communes. Accueillir les administrés disposer de compétences en urbanisme, s'occuper de l'état civil. Avoir une expertise budgétaire, juridique ou en marche en matière de marchés publics. Organiser les élections où le recensement parfois gérer les ressources humaines, préparer les conseils municipaux rédiger les procès-verbaux et les 10 les délibérations, les secrétaires de mairie sont polyvalente et confine au couteau suisse. Ce sont les maires qui en parlent le mieux. Ils attendent de pouvoir travailler en symbiose avec la secrétaire de mairie et combien d'entre eux se sentent complètement démunis quand ses chevilles ouvrières communal viennent à manquer. Et ce d'autant que la dématérialisation des procédures s'accroît, que les trésoreries se sont éloignés distant dans parfois les Liens avec le percepteur que les intercommunalités se sont agrandis. Compliquant les difficultés pour les plus petites communes de se faire entendre que l'État abandonne parfois ses propres missions, celle d'assurer l'égalité républicaine l'égalité territoriale par exemple mais se fait plus intrusif et plus procédurier à l'égard des communes. J'ai été interpellée par des élus de la Seine Maritime, parce qu'il manquait une cinquantaine de secrétaire de mairie dans mon département, il y a un peu plus d'un an de cela, il en manque désormais une centaine d'après l'Association des maires et près de 2000 à l'échelle du pays, de nombreux secrétaires de mairie nous font aussi régulièrement par des soucis qu'elle rencontre et surtout de leurs nombreuses propositions pour reconnaître et rendre attractive leur profession. Je sais que chacun de nos collègues ici en est pleinement conscient comme le sont les associations d'élus qui travaille depuis plusieurs mois maintenant à des propositions permettant de revaloriser ce métier. 30% des secrétaires de mairie sont appelés à partir en retraite d'ici 2030. Il faut donc impérativement recruter de nouvelles de nouveau. Faute de quoi le fonctionnement de nos communes. Les services qu'elles rendent au quotidien les projets les réalisations attendues par les habitants en pâtiront. Se pencher sur le sort. Le sort des secrétaires de mairie. C'est une question de justice à l'égard de celles et je dis volontairement celle depuis le début de mon propos, car ce sont des femmes pour 94% d'entre elles qui exerce ce métier mal connu, mal considéré. Mal rémunérés, c'est aussi un enjeu en matière de services publics de proximité de maillage territorial et même un peu de cohésion nationale. Nous constatons actuellement un nombre de démissions jamais égalée parmi les élus locaux. Je n'en tire pas de conclusions trop hâtives mais sans doute que le sentiment d'abandon que vivent les élus de nos petites communes comme le vif d'ailleurs, nombre de nos concitoyens n'est pas étranger à ce phénomène. Ils ont besoin d'être accompagnés dans l'émission qui se complexifie besoin d'être soutenus dans un engagement qui peut parfois sembler ingrat besoin que le temps et l'énergie qu'ils consacrent à leur mandat trouvent toute leur utilité toute leur efficacité et de ce point de vue les secrétaires de mairie à compétences leur rôle au côté des mères de leurs adjoints de l'ensemble des conseillers municipaux sont décisifs. C'est un peu de l'existence même de nos communes qui se joue, nos communes au coeur de la République n'existerait pas sans les élus qui les font vivre en s'appuyant sur les secrétaires de mairie, ce sont ceux-là mêmes vers lesquelles se tournent même le plus jupitérien des présidents à chaque nouvelle crise. Je souhaite remercier mes collègues du groupe communiste citoyen républicain écologiste d'avoir pris l'initiative de mettre cette proposition de loi dans l'une de ses niches remercier aussi la commission des lois, son président ça rapporteur qui se sont emparés avec bienveillance du sujet sur le plan de la formation en premier lieu avec la volonté de mettre en place une formation solide pour les secrétaires de mairie, avec l'instauration d'une formation obligatoire commune à l'ensemble d'entre elles dans l'année de leur prise de poste, c'est une demande de leur part quand elles ont trop souvent dû se former sur le tas ou bénéficier de l'apport de leurs prédécesseurs. Ce qui est toujours appréciable mais pas forcément suffisant. C'est aussi un souhait des élus locaux des maires en particulier car leur confiance dans les secrétaires de mairie s'appuie avant tout sur les compétences de celle-ci. Sur le plan de la promotion interne ensuite afin de leur offrir des perspectives de carrière, qui font trop défaut aujourd'hui. L'établissement de listes d'aptitudes par l'autorité territoriale ou le cas échéant, le président du Centre de gestion devra ainsi mieux tenir compte de l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie, chacun sait que l'accès aux catégories supérieures de la fonction publique, par voie de concours de promotion interne a un impact concret sur le niveau de rémunération pour faire face aux difficultés de recrutement de recrutement qui se posent, enfin avec urgence avec un élargissement de la possibilité de recourir aux contractuels pour pourvoir les postes de secrétaire de mairie dans les communes de 1000 à 2000 habitants en cas d'absence de titulaire mais cette proposition. La loi de loi n'est, n'épuisera pas à elle seule, loin de là, la totalité des sujets liés au métier de secrétaire de mairie beaucoup sont d'ordre réglementaire et donc de votre responsabilité. Monsieur le Ministre et je voudrais vous interpeller très solennellement. Nous voudrions ainsi que soit poursuivi le chantier de la formation initiale et continue et que des mesures soient déployés pour faire connaître faire happer apprécié rendre accessible et lisible ce bel et indispensable métier. Le statut des secrétaires de mairie a changé avec l'extension du Cadre d'emplois spécifiques reconnu de catégorie A en 2001 et il n'y a plus aujourd'hui de Cadre d'emplois particulier qui soient rattachés des agents titulaires de la fonction publique territoriale des différentes catégories A, B et C peuvent exercer ce métier. Or aujourd'hui les secrétaires en poste appartiennent essentiellement à la catégorie C avec des salaires nettement insuffisant face aux responsabilités qui leur incombent la technicité dont elles doivent se doter la polyvalence des tâches qui rythment leur quotidien. Nous voudrions que vous entendiez que malgré la bonification indiciaire augmenté de 15. Accordés au secrétaire de mairie, il y a maintenant un an, ce qui représente un gain brut de 70 euros par mois. Les secrétaires de mairie sont insuffisamment rémunéré au regard de leur mission. On ne créera pas le choc d'attractivité nécessaire en les maintenant à des salaires à peine plus élevés que le SMIC. Nous voudrions que vous pères soviets que les communes font face elle aussi à une redoutable inflation à la crise énergétique et que leurs finances sont compliquées. C'est un appel, vous l'aurez compris, à mieux compenser la revalorisation du point d'indice décidiez, il y a quelques mois à mieux compenser celle qui doit voir le jour en direction des secrétaires de mairie, notamment avec la délégation aux collectivités territoriales dont je salue la présidente avec l'ensemble de nos collègues, nous allons continuer de travailler sur cette indispensable revalorisation du métier des secrétaires de mairie. C'est nécessaire pour nos petites communes mais nous espérons Monsieur le Ministre que vous mesurez l'urgence face à laquelle nous sommes et vous prendre et que vous prendrez les décisions qui s'imposent. En tout cas compter sur nous pour ne rien lâcher sur ce sujet là aussi je vous remercie. Merci cher collègue là. Parole est maintenant à Madame, Catherine Di Folco, rapporteur de la commission des lois pour 10 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le président de la commission des lois, chers collègues, nous examinons la proposition de loi déposée par Céline Brulin, et ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste visant à revaloriser le statut de secrétaire de mairie et je les remercie sincèrement pour cette initiative. Comme l'a rappelé son auteur. Cette proposition de loi a pour objectif d'esquisser des réponses face au manque d'attractivité dont souffre aujourd'hui le métier de secrétaire de mairie. Il s'agit d'une question essentielle à la fois pour les communes de moins de 2000 habitants dont le fond le bon fonctionnement dépend largement du travail considérable accompli par ses agents. Et pour les secrétaires de mairie elles-mêmes ou eux-mêmes qui sont aujourd'hui insuffisamment reconnue. Faute de mesures concrètes et rapides et compte tenu de la pyramide des âges, la pénurie de secrétaire de mairie à la cas à laquelle font face aujourd'hui la quasi-totalité des mères ne peut que s'aggraver. Il est donc urgent de répondre aux besoins légitimes de reconnaissance de ses agents indispensables à la bonne gestion municipale en milieu rural et de leur garantir entre autres une rémunération et des conditions de travail à la hauteur de leurs responsabilités. La commission des lois partage donc pleinement l'objectif de la présente, proposition de loi. Afin de garantir la nature législative de ces dispositions et de les rendre pleinement opérationnel. Elle a apporté un certain nombre de modifications au texte initial. En premier, la commission a tout d'abord considérer que la création d'un statut d'emploi de secrétaire de mairie ne serait guère opportune en effet un tel statut ne permettrait pas d'offrir des perspectives de carrière améliorée au secrétaire de mairie ni ne constituerait un facteur particulier d'attractivité. En outre, un statut d'emploi serait incompatible avec la spécificité du métier de secrétaire de mairie qui comme vous le savez peut être exercée par des fonctionnaires relevant de 4 Cadre d'emplois différents et trois catégories hiérarchiques distinctes. En tout état de cause, si la création d'un statut d'emploi relève de la loi, les conditions d'accès à un tel statut relève quant à elle du règlement de même que la création éventuelle d'un cadre d'emploi et le nom choisi pour celui-ci et donc pour toutes ces raisons, la commission a supprimé l'article 1er. Ensuite, la commission a souhaité conforter la formation des secrétaires de mairie qui est essentielle au regard de la variété des missions exercées et de la technicité des compétences requises. L à substituer aux dispositions initiales des articles 3 et 4, l'introduction d'une formation initiale obligatoire propre à ses agents. L'objectif est de que chaque secrétaire de mairie dispose dès sa prise de poste, des outils adaptés pour exercer ses missions. Nous avons en effet. Combien il est difficile au secrétaire de mairie de suivre des formations, même de quelques jours par manque de temps par l'éloignement géographique du lieu de formation et surtout en raison de la quasi-impossibilité à se faire remplacer en leur absence. Par ailleurs, la commission a estimé nécessaire de garantir les perspectives d'évolution de carrière au secrétaire de mairie, par la voie de la promotion interne au delà des dispositions réglementaires qui existent déjà. Elle a donc modifié l'article 5 de la proposition de loi pour y inscrire la prise en compte obligatoire de l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie pour l'établissement des listes d'aptitudes par les présidents des centres de gestion. Enfin, la commission a souhaité offrir une réponse aux difficultés de recrutement que rencontrent les communes de moins de 1000 habitants. Elle reconnaît d'une part que ces difficultés sont de nature budgétaire toutefois elle a considéré que la création d'un fonds de soutien local financé par l'État, telle que le proposait l'article 6 de cette proposition de loi ne serait pas adaptée. En effet, les communes ont vocation à disposer de ressources libres d'emploi plutôt qu'à recevoir des dépenses liées au recrutement d'agents. Un soutien financier de l'État, c'est l'occasion de le rappeler l'autonomie financière dont ont besoin les communes ne saurait passer par une compensation mais doit passer par une fiscalité adaptée, ainsi que par l'indexation de la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation. En outre, la création d'un nouveau fonds renforcerait la complexité des relations financières entre l'État et les collectivités territoriales. C'est pourquoi la commission a supprimé les articles 6 et 7. Afin de faciliter le recrutement de secrétaires de mairie pour par les communes de moins de 2000 habitants. Elle a en revanche ouvert aux communes comptant entre 1000 et 2000 habitants la possibilité de recruter des agents contractuels. Pour les emplois de secrétaire de mairie à temps complet. Je précise qu'aujourd'hui elles peuvent déjà le faire pour les emplois à temps non complet. La commission des lois vous propose donc d'adopter cette proposition de loi ainsi modifiée qui offrent des ajustements et des précisions de nature à améliorer la formation et et les perspectives de carrière des secrétaires de mairie d'une part et à faciliter le recrutement par les communes. D'autre part. Tout le monde s'accordera je pense sur le fait qu'il s'agit d'aménagement bienvenue mais qui ne pourront régler à eux seuls la question complexe de l'attractivité du secrétaire de mairie madame brûlant là déjà évoqué. Si le législateur ne sont me semble être allé au bout de sa compétence sur le sujet. Il revient désormais au pouvoir exécutif de travailler à des voeux évolution concrètes j'invite donc le gouvernement à se saisir de cette question urgente pour revoir, entre autres, les règles relatives à la rémunération et à la carrière des secrétaires de mairie. Vous le savez les instruments de rivaliser revalorisations salariales qui existe aujourd'hui présente des limites qu'il s'agisse de la mise en oeuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel, ou de la valorisation de la nouvelle bonification indiciaire la NBI. Je conviens que l'attractivité d'un métier ne se résume pas à sa fiche de paye. Mais comment s'étonner du manque d'attractivité du métier de secrétaire de mairie, comme beaucoup d'autres métiers de la fonction publique territoriale d'ailleurs lorsque la rémunération horaire d'un secrétaire de mairie adjoint administratif principal de première classe qui compte déjà 32 ans d'ancienneté dans la fonction publique territoriale et de 13 75 euros soit seulement de 68 euros de plus que le SMIC brut, on peut se poser des questions effectivement. Dans ces conditions, il est primordial. Monsieur le Ministre que vous accordiez une attention toute particulière à la situation des secrétaires de mairie dans le cas des travaux portant sur l'accès, les rémunérations et les parcours professionnels dans la fonction publique chantiers que vous venez de lancer. Enfin, les difficultés à connaître le métier de secrétaire de mairie et à moderniser l'image qu'il renvoie auprès des jeunes Iraniens ration met en lumière la nécessité de mener aussi une réflexion de fond sur les moyens d'améliorer la visibilité des métiers de la fonction publique territoriale. Il est essentiel que les employeurs publics et notamment les employeurs territoriaux se dote d'une véritable public de. Une véritable politique de communication qui donne à voir l'extrême variété des carrières à mener donc Monsieur le Ministre, vous l'aurez compris, la balle est dans votre camp. Et je vous remercie pour votre attention. Merci cher collègue. Hé bien vous y êtes invités doublement Monsieur le Ministre, la parole est à monsieur Stanislas Guerini Ministre de la transformation et de la fonction publique. Je prends Je prends la balle au bond. Madame la rapporteure. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois. Madame la rapporteur, madame la sénatrice Céline Brulin. Mesdames, et messieurs les sénateurs, vous avez choisi, aujourd'hui, d'examiner un texte qui porte sur un métier essentiel. Celui de secrétaire de mairie, coeur battant des communes en particulier des communes rurales bras droit des mères pilier au quotidien pour les habitants. Quand on est ministre de la fonction publique. Je crois qu'on peut dire qu'il y a pas une semaine sans échanger sans parler de ce beau métier de secrétaire de mairie parfois avec les élus locaux évidemment parfois directement avec des secrétaires de mairie je pense. Par exemple à cette vie JBL qui a lancé un collectif de secrétaire de mairie dans le Gers qui réunit aujourd'hui plus de 2000, secrétaire de mairie. J'ai mesuré. À chaque occasion à quel point il est bien plus souvent elle vous l'avez rappelé, sont un rouage essentiel entre les élus municipaux et la population. Budget. État civil. Urbanisme bonne marche des services publics du quotidien. Je ne serai pas plus long, on pourrait évidemment et vous l'avez excellemment faire allonger ici la liste Non sans un certain paradoxe face à ces exigences. C'est l'un des métiers de la fonction publique territoriale dont le profil ou les qualifications requises sont les moins bien défini. C'est probablement aussi. L'un de ceux les plus confrontés à l'enjeu de meilleure reconnaissance en terme de rémunération. Et ce malgré. Vous l'avez rappelé également l'effort accompli en 2022 pour revaloriser leur NBI. Mais avec trop souvent encore l'absence de régime indemnitaire. J'ajoute que ce sont. Des conditions d'emploi qui sont rendues compliquées par le partage des fonctions entre plusieurs employeurs, là aussi vous l'avez rappelé dans les plus petites communes. Autant de facteurs. Qui jouent négativement sur l'attractivité de ce métier, alors même que la démographie va accentuer encore les tensions de recrutement. Le constat lucide conduit à dire que d'ici huit ans. Ce sont un tiers des secrétaires de mairie qui seront partis à la retraite. J'ai eu souvent l'occasion de le dire. Les premières maisons France service ce sont les guichets des communes. Alors disons-le simplement, une secrétaire de mairie qui part à la retraite et qui n'est pas remplacé. C'est comme si on fermé de maison Francis. Nous devons agir. Sans attendre pour rendre ce métier plus attractif. Il est vital pour l'avenir de la commune et de nos services publics et je sais que c'est une préoccupation partagée ici au Sénat et au sein du gouvernement. Alors je tiens dans ces conditions, a salué le débat que vous nous permettait d'avoir aujourd'hui sur l'avenir de ce métier de secrétaire de mairie. Je souhaite d'abord relevé de points. D'abord madame la sénatrice, je relève tout d'abord que dans votre proposition, vous avez considéré la fonction de secrétaire de mairie comme un métier à part entière. Je trouve cette approche pertinente. Au-delà de ses seules caractéristiques statutaire ou catégoriels. Elle nous permet de prendre en compte la globalité. Des conditions d'emploi, de formation, de parcours. Quelle que soit l'appartenance statutaire des agents concernés. Je vous le dis, sans ambiguïté, vous me trouverez toujours défenseur du statut. Je suis convaincu qu'il reste un cadre adapté face au défis que le service public doit aujourd'hui relever. Je crois que personne ne soupçonnera le groupe communiste de vouloir et porter atteinte, mais je souhaite remercier les auteurs de ce texte pour leur pragmatisme qui nous permet aujourd'hui un échange très concrets sur cette approche métier. Mon second point d'intervention fait écho au débat que vous avez eu en commission très simplement madame la rapporteure pour. Confirmer que l'essentiel des dispositions envisagées relève davantage du Champ réglementaire. Cela n'invalide en rien la pertinence des questions soulevées, nous pourrons en toute hypothèse mettre au crédit de ce débat, que celui-ci nous pousse utilement à agir. Et donc je poursuivrai les travaux que nous avons initiée avec les employeurs territoriaux. L'Association des maires de France, l'association des maires ruraux de France ou encore la Fédération nationale des centres de gestion. Donc je partage une large part des propositions. Je voudrais à cet égard partager avec vous les orientations que nous poursuivrons avec ma collègue Dominique Faure Ministre délégué en charge des collectivités territoriales et de la ruralité. Comme votre proposition de loi le suggérait. Nous souhaitons agir sur plusieurs axes. Le recrutement, les compétences, les parcours et rémunération. Le recrutement d'abord. Vous souhaitez élargir le recrutement de contractuels pour les communes jusqu'à 2000 habitants. J'y suis favorable. Ce sera effectivement un outil supplémentaire à la main des maires mais disons-le clairement, il ne résoudra pas tout. C'est pourquoi vous m'y avait appelé je réponds à cet engagement nous nous mobiliserons pour mieux faire connaître ce métier auprès du grand public est démultiplié le vivier de candidats et de candidates potentielles. Cela passe notamment par un partenariat que j'encourage de mon ministère encourage entre Pôle emploi, le Cnfpt, les centres de gestion pour promouvoir les offres de recrutement et développer des formations pour les demandeurs d'emploi. Peut être aussi c'est une question que vous avez mis au débat. Faudra-t-il donner un autre nom à ce métier. Pour qu'ils puissent mieux traduire ses missions. Je suis favorable, je n'ai pas encore David définitivement arrêtée sur le nom même et je suggère que cette nouvelle dénomination soit travailler avec les secrétaires de mairie elles-mêmes ainsi qu'avec les employeurs territoriaux. Je proposerai également et je pense que nous devons mener une réflexion sur cette idée là que cette fonction puisse être occupés par des profils plus divers issus de toutes les filières au-delà même des seules filières administratives. Ce sera une occasion d'élargir le vivier de recrutement, posons-nous la question des agents de guichet France services peuvent devenir par exemple demain des secrétaires de mairie pour ne prendre qu'un exemple. Plus largement. Et je crois que sans tabou, on doit aussi réfléchir à l'hypothèse que vous avez mis au débat de la fonctionner actions ses employes secrétaire de mairie dans les communes de moins de 2000 habitants. Il nécessite un travail législatif plus approfondi, mais nous ne devons pas écarter cette réflexion je veux enfin apporter des réponses à la problématique des temps non complet et permettre de façon mieux cadrer aux intercommunalités et au centre de gestion de recruter des agents qualifiés pour les mettre à disposition des mairies afin d'exercer les fonctions de secrétaire de mairie. Sur les compétences ensuite. Il me semble essentiel, je crois, à vous entendre que cette une idée partagée de redéfinir le socle de compétences requis pour être secrétaire de mairie. C'est l'une des priorités auxquelles nous devons nous atteler avec les représentants des employeurs territoriaux sur cette base souhaite la mise en place de formations adaptées. D'abord une formation qu'on pourrait qualifier de formation, de qualification. Pour les agents qui candidat très et qui ne disposerait pas de ce socle de base. Je le dis là aussi clairement. Le niveau de responsabilité exercée par un secrétaire de mairie me paraît relever au moins de la catégorie B. Mais ça doit pas empêcher de recrutement comme aujourd'hui d'agents de catégorie C mais il faut alors que ceux-ci acquièrent le niveau de qualification requis. Grâce à cette formation qu'on pourrait qualifier de formation, de qualification. Il convient par ailleurs de mettre en place une formation qu'on pourrait appeler formation de professionnalisation modulée en fonction du parcours antérieurs des titulaires. Cela rejoint pour partie l'article 4 de votre proposition. Enfin. Nous devons agir sur les rémunérations et les parcours. Si nous. Fonctionne Allyson l'emploi de secrétaire de mairie. Il nous faudra pour en déterminer le niveau de rémunération et sa progression, prendre en compte tant la taille des communes que la pluralité des viviers. Il y a donc place à définir des solutions innovantes en la matière. Je me dois au passage de rappeler que s'agissant du résume indemnitaire les textes actuels offrent d'ores et déjà aux maires des marges importantes. C'est un levier d'attractivité immédiatement mobilisables. Même si j'ai conscience que cela vous l'avez mentionné également représente un coût salarial. Mais peut-être que la mutualisation de l'emploi de secrétaire de mairie entre plusieurs petites communes peut aider aussi parfois et faire face. Enfin, le parcours de carrière devraient être encouragés à tous les niveaux. Que ce soit pour valoriser la qualification acquise par un agent de catégorie C exerçant l'emploi de secrétaire de mairie. Ou pour favoriser grâce à l'exercice de ce métier. L'accès à des emplois ou à des corps supérieur. Je comprends que c'est dans cet esprit que les proposé votre article 5 même si je n'en partage pas tout à fait la formulation. On a un moment où nous cherchons plutôt à alléger les quotas. Qui encadre les promotions, cela fait partie des objectifs que je recherche aussi. Alors voilà. Autant de pistes de travail qui s'inscrivent en cohérence avec le chantier d'ensemble sur l'attractivité de la fonction publique dont j'ai fait ma priorité. J'ai partagé les orientations avec les partenaires sociaux et les représentants des employeurs territoriaux. Autant de propositions que j'approfondir. Dès les prochaines semaines avec eux sur la base, sur la je serais heureux de poursuivre le travail autant que nécessaire avec les parlementaires. Mesdames, et messieurs les sénateurs. C'est donc dans cet esprit et avec cette volonté que le gouvernement porte aujourd'hui un avis de sagesse sur votre proposition de loi qui présente des premières avancées. Je crois qu'on peut le dire, éclaire le chemin qu'il nous faut poursuivre. Je vous remercie. Très bien, merci Monsieur le Ministre, dans la suite de la discussion générale. La parole est immédiatement madame Cécile Cukierman. Pour le groupe CRCE pour cinq minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cela a été dit, le métier des secrétaires de mairie si les peut être peu connu du grand public il est énormément connu apprécié et fondamental auprès de tous les élus locaux. Si nous pouvions résumer en quelques mots le travail de ses secrétaires de mairie, nous pourrions dire qu'elles sont la clef de voûte du Maillon communal de ce dernier service public qui existe dans nombre de nos communes rurales. Je dit-elle en parlant de ses secrétaires de mairie car aujourd'hui ce métier, ce sont 94% des des femmes qui l'exerce. Elles doivent disposer d'ailleurs et cela a déjà été dit de savoir-faire dans de nombreux domaines domaine filon sinon pardon domaine rédactionnel technique également des domaines dans la qualité humaine de la relation avec des administrés des administrés dans tous nos territoires qui sont de plus en plus exigeant. Une rigueur également dans une société où la judiciarisation se développe et où toute erreur peut avoir des conséquences très importantes pour la commune. Pour le maire et l'ensemble du conseil municipal. Pour autant ce socle de base et vous y avez fait référence Monsieur le Ministre est en constante évolution ce métier s'est profondément transformé au cours de ces dernières années parce que. La politique communale c'est même profondément transporté m'a transformé ma collègue Céline Brulin le rappelait le poids aujourd'hui des intercommunalités et nous avons tous en tête des secrétaires de mairie qui passant d'une commune à l'autre n'étant pas dans les mêmes intercommunalités rajoute de la complexité à ce métier. Nous avons également tous en tête. La dématérialisation décidé fait pour simplifier et qui dans de nombreuses communes rajoute en forte complexité à ce métier et à son exercice, alors je l'ai dit, ce sont ces secrétaire de mairie qui gère aujourd'hui dans toutes les communes, les questions de l'urbanisme, des projets d'aménagement de la recherche de financements de plus en plus nécessaire et en 10, indispensable pour pas satisfaire les investissements dans nos communes. Ce sont elles qui reçoivent les usagers et disons-le, ce sont elles qui bien souvent font beaucoup plus que simplement les propres missions qui devraient être les leurs. Leur statut n'est pas à la hauteur de ce qu'elle représente au quotidien. Leur rémunération sont faibles 62% exercent à temps non complet 24% partagent leur travail sur 3 communes pour obtenir et madame la rapporteure la rappeler à la fin du mois un salaire. Convenable entre guillemets, 60% sont des agents de la catégorie C et ne permettent pas pour beaucoup de pouvoir bien en vivre aujourd'hui ce sont plus de 1900 postes qui demeure à pourvoir le métier manques inévitablement d'attractivité. D'autant plus que dans les années qui viennent et d'ici à 2030 un tiers des postes aujourd'hui effectués devront partir à la retraite. Il y a donc à la fois, urgence, urgence tout d'abord à satisfaire à ces postes non pourvus, il y a urgence à anticiper et c'est pour cela que nous avons proposé à travers cette proposition de loi notamment un travail sur les enjeux de formation parce qu'il y a besoin d'anticiper, d'ores et déjà les vacances de postes à venir si l'on ne veulent pas qu'elles viennent se rajouter à celles existantes et il y a effectivement une véritable réflexion à avoir sur la rémunération parce que si l'argent ne fait pas le bonheur et ne fait pas tout, il y contribue quand même fortement et on s'en rend compte, en tout cas sur un certain nombre de postes. Dire cela s'est également rappelé. Et et nous avons avec beaucoup d'humilité déposée en mars 2022. Cette proposition de loi parce que. Fortement sollicité les uns et les autres, je l'ai déjà dit il y a ce besoin d'améliorer ce statut. Tout n'est pas du ressort du travail législatif, nous en sommes pleinement conscients. Il y aura donc un travail réglementaire et Monsieur le Ministre, c'est aussi pour cela que nous vous interpellons il y aura très certainement un véritable travail local à avoir, et je crois que il n'y a pas à décider ici s'il faut demain mutualisés à l'échelle intercommunale mutualisés à l'échelle départementale ou à je ne sais quel autre échelle, ces métiers là il y aura en tout cas besoin d'avoir de véritables réflexions pour réfléchir effectivement localement en fonction de nos territoires en fonction de la taille des communes en fonction des distances y compris entre celle-ci a la capacité à mutualiser plus ou moins certains postes pour à la fois satisfaire en matière de compétence satisfaire en matière de salaire. Ses différents métiers. En tout cas, et en l'état sans surprise nous voterons cette proposition de loi, je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est maintenant madame Nathalie Goulet, pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. c'est le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le président de la commission des lois. Madame la rapporteure. Il convient évidemment de remercier l'auteur de cette. Proposition et le groupe. Qui l'a mise à l'ordre du jour. Je pense que c'est une excellente idée à la texte elle atteste de notre proximité avec les secrétaires secrétaires de mairie qui sont les chevilles ouvrières les couteaux suisses. Enfin, nous faisons tous évidemment le même constat. Nous les avons au téléphone régulièrement et la description qu'qui a fait Céline Brulin tout à l'heure. À la à la tribune. Oh, je crois qu'on pourrait évidemment. Tous le faire ici. On sait à quel point leur présence est indispensable

évidemment se reposent sur leurs. Compétences et d'ailleurs. Pas un hasard si elles reçoivent régulièrement des mais des médailles. Régionales, départementales et communales qui sont l'espèce de Légion d'honneur des des et on associe les personnels communaux. Ils, ils font équipe et donc tout ça contribue évidemment à reconnaître leurs mérites, mais pas seulement. Donc belle unanimité des constats assistante. Évidemment de mairie mais aussi des des citoyens, surtout dans les zones rurales et elle reste finalement bien souvent le seul élément d'humanité sur le diktat de la dématérialisation, vous avez parlé des maisons France service mais les secrétaire de mairie les remplace évidemment et effectivement ce que vous avez proposé. D'interopérabilité, si j'ai bien compris, entre les maisons France service et les secrétaires de mairie serait effectivement une solution intéressante. Le manque d'attractivité de la fonction. Correspond aussi à un moment ou jamais. Le nombre de démissions d'élus n'a été aussi important et je pense que là il y a il y a un phénomène convergents qui est probablement liée. Pardonnez-moi l'expression mais oh diarrhée législative et réglementaire et et aux difficultés d'appréciation et d'interprétations administratives à une espèce de rigueur administrative dont notre pays a aussi le secret. Les secrétaires de mairie sont souvent isolés peut être promouvoir le travail en réseau, les centres de gestion le s'éveille aux formations. Mais le malaise demeure et le débat reste utile. Alors j'ai déposé un amendement d'appel. Vous avez fait. Allusion les uns et les autres au nom. Effectivement, secrétaire de mairie n'peut-être pas exactement le terme idoine collaborateur du maire non plus parce que le maire correspond. À une autre fonction et la secrétaire de mairie et là pour la mairie et les concitoyens. Je pense qu'il faut évidemment engager une réflexion, je vous propose que nous la menions ensemble. Sans avoir recours au cabinet McKinsey. Et donc je crois que là on a, on a une une une une solution qu'il faut évidemment trouver ensemble et puis on a parlé, on a parlé de qualification tout à l'heure. On a On a parlé de de d'améliorer les salaires mais là aussi il faut faire attention parce que dans le Mikado. De la fonction publique territoriale. Et des grades. De la politique. Territoriale. Il faut aussi maintenir une différence avec ceux de nos agents qui eux passent des concours difficiles, donc c'est, c'est assez compliqué et je crois que la réflexion évidemment s'impose donc. Ce texte est un signal, il faut évidemment pas manqué de poursuivre. La démarche et évidemment nous voterons avec enthousiasme les dispositions restant après l'examen en commission des lois. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant Madame Maryse Carrère pour le groupe RDSE pour cinq minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteur, madame. L'auteur de la proposition de loi. Monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues. Il y a très longtemps, l'instituteur du village faisaient souvent office de secrétaire de mairie. L'intégration des communes rurales au sein de structures supra-communal et l'évolution des lois et de la réglementation en considérablement bouleversé la nature des tâches des années 60. Aujourd'hui ses agents essentiellement des femmes constituent un maillon indispensable au bon fonctionnement des petites communes principalement en milieu rural et plus la commune est petite, plus leur rôle est décisif. Elles mettent en oeuvre les décisions du conseil municipal gère les ressources humaines, participe à l'élaboration du budget rédiger les documents administratifs et sont les interlocuteurs privilégiés des usagers agent dévoué sur lesquels les mères, elles s'appuient quotidiennement. Elles sont devenues de vrais couteaux suisses comme elle aime à se définir. Mais ce métier est intention et bien que les élus locaux redouble d'efforts pour susciter des vocations, il attire de moins en moins de candidats et la pénurie va s'aggraver avec les nombreux départs en retraite. Comme vous l'avez rappelé. Monsieur le Ministre, environ un tiers des secrétaires de mairie ça se rend leur activité dans les huit l'année prochaine. Les raisons de cette désaffection sont bien connus. Rémunérations faibles exigences de compétences variées fortes responsabilités et obligations pour beaucoup de cumuler des postes dans plusieurs petites communes pour pas parvenir à un temps plein. Sans parler de la formation et de l'évolution professionnelle, qui ne sont pas suffisamment accompagné le métier concentre à lui seul les difficultés de la fonction publique territoriale. Cette vague de départs pousse les maires à recruter des profils qui n'ont pas forcément de compétences territoriales ou à procéder dans l'urgence à des. De secrétaire de mairie ce qui alourdit encore plus leur charge de travail. En novembre 2021, Amélie de Montchalin, alors ministre de la transformation de la fonction publique promettait plusieurs évolutions dans un souci de valorisation et de reconnaissance du mythe heure. Nominations de la fonction. Un secrétaire général de mairie une revalorisation indiciaire un accès facilité aux contrats santé et prévoyance ainsi que des améliorations, s'agissant de la formation. L'idée était intéressante. Pourtant, force est de constater que l'on n'a pas beaucoup avancé sur le sujet. En effet, une seule mesure a été mise en oeuvre la nouvelle bonification indiciaire la NBI a été revalorisé de 15 points au 1er mars 2022 pour les secrétaires de mairies des communes de moins de 2000 habitants. Cette mesure est toutefois limité comme l'a rappelé notre rapporteur puisqu'elle ne concerne pas les agents contractuels et toutes les communes ne semble pas avoir pris l'arrêté permettant sa mise en place. La réponse nous semble donc bien insuffisante face aux défis qu'il nous faut relever. Le Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales organisée en septembre dernier, un colloque intitulé secrétaire de mairie espèce menacée de la territoriale ou clé de voûte du bloc local au XXIe siècle. Tout est dit. C'est pourquoi je salue l'initiative de nos collègues du groupe CRCE ainsi que le travail de notre rapporteure le texte que nous examinons ce matin entend répondre à un impérieux besoin sur nos territoires et relancer l'attractivité de ce métier mal connu et mal reconnu. Je me félicite notamment de l'introduction d'une formation initiale obligatoire à propres secrétaire de mairie. Adaptées à la spécificité de leur mission, elle sera dispensée par le Cnfpt, dans l'année qui suit la prise de poste, c'est une excellente chose. La proposition de loi telle qu'elle résulte des travaux de notre commission met également en place les moyens de leur garantir des perspectives d'évolution de carrière. Enfin notre commission a introduit une nouvelle disposition pour permettre aux communes de 1000 à 2000 habitants de recruter des agents contractuels pour les emplois de secrétaire de mairie. Cette disposition fait débat, y compris au sein du groupe RDSE pour autant pour nous priver ces communes de la possibilité de recruter un agent contractuel sur un emploi de secrétaire de mairie à temps complet, je ne le crois pas. Mais prenons garde quand même à préserver. Le, l'évolution dans la fonction publique territoriale. Monsieur le Ministre, vous avez lancé le 1er février dernier, les travaux sur l'accès les parcours et les rémunérations dans la fonction publique. J'espère que cette réforme d'ampleur sera l'occasion de relancer l'attractivité du métier de secrétaire de mairie. Avec cette proposition de loi que nos collègues vous nous propose, nous ouvrons cette voie et nous voterons cette proposition à l'unanimité du groupe RDSE. Je vous remercie. Merci. Cher collègue, la parole est maintenant Monsieur Cédric Vial pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes.

Monsieur le président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La proposition de loi que nous étudions aujourd'hui en hémicycle a le mérite de nous permettre. De pouvoir évoquer cette problématique que nous connaissons tous dans nos territoires, celui du métier de secrétaire de mairie des difficultés afférentes à l'exercice de ses missions et à l'attractivité de ses fonctions. Il s'agit pourtant d'un beau métier. Un métier complet, polyvalent au service du public, c'est un métier qui a du sens, un métier où l'on trouve des solutions. Bref, un métier utile. Pourtant ces agents de l'ombre qui sont souvent la dernière porte accessible des services publics dans nos territoires ruraux. Ces agents qui sont sur tous les fronts administratif, juridique, politique stratégique mais aussi social. Ces agents qui doivent souvent cumuler des postes. Dans différentes mairies pour espérer avoir un temps plein. Et surtout ses agents qui manque dans nos territoires, à tel point que ce sont les maires qui doivent dans de nombreuses mairies cumuler à la fois les fonctions de maire et le métier pourtant très technique de secrétaire de mairie. Aujourd'hui, en mars 2003, 2023 environ 2000 postes de secrétaire de mairie était publié sur le site emploie territoriale. Il faut se rendre à l'évidence ces postes n'attire plus. Et ce n'est qu'un début. Lorsque nous observons qu'un quart des agents en poste ont plus de 58 ans et que 60% ont plus de 50 ans. Nous avons d'ores et déjà qu'un tiers des secrétaires de mairie vont partir à la retraite dans les 6 prochaines années. En l'espace de 20 ans c'est pas son été fortement impactée par l'évolution de nos institutions locales notamment avec le transfert des compétences de l'État en direction des collectivités. Le secrétaire de mairie paye le prix fort du désengagement de l'État dans les territoires auparavant lorsque ses agents avaient un doute ou une question il pouvait faire appel aux services de l'État de la DDT de la trésorerie. Aujourd'hui, ils doivent se débrouiller, le plus souvent seuls et le sentiment de solitude ne fait que s'accentuer. De réforme en réforme. La bureaucratie frénétique avec une des législations débordante et une réglementation prolifique rend la mise en oeuvre de projets ou d'action impossible si vous n'êtes pas expert les secrétaires de mairie doivent-ils être expert en tout. Nous savons tous ici, que ce n'est pas possible. Nous aurions aussi pu imaginer que la création des intercommunalités et leur renforcement allait pouvoir aider les territoires mais il ressort des retours de terrain que cela s'est traduit négativement pour les secrétaires de mairie le partage de responsabilités entre la commune et les EPCI. N'est pas si clair qu'on veut bien des fois bien le croire. L'intégration d'une commune. Au sein d'une intercomités se traduit souvent par de nouveaux process de nouvelles charges de travail avec un surcroît de développement d'un sentiment de déclassement ou de dépossession pour nos secrétaires de mairie. Toutefois, ce n'est plus l'heure des constats, mais celui de l'action. La proposition que loi que nous étudions aujourd'hui à l'initiative de nos collègues du groupe communiste constitue un début de réponse. Et nous la voterons comme je l'espère. Large majorité du Sénat car nous voyons tous dans nos territoires des secrétaires de mairie Abou usés et désabusés. Ou encore des maires inquiets de voir des recrutements infructueux pour le poste de leur secrétaire de mairie sans lesquels ils ne peuvent pas exercer la plénitude de leurs fonctions et donc de leur mandat. Toutefois, je crains que les secrétaires de mairie ne soient déçus car cette proposition de loi ne répond malheureusement pas la totalité des enjeux qui se posent à nous. Et j'en profite pour saluer à la fois le travail de la commission des lois de sa rapporteur hein Catherine Di Folco et le sens de responsabilité de ses auteurs Céline Brulin, Cécile Cukierman et Michelle. Gréaume qui ont permis pardon d'aborder ce texte et de le rendre acceptable et et consensuel, grâce à un travail collaboratif et transpartisan dont le Sénat a désormais.

Le travail amorcé aujourd'hui sur le plan législatif avec cette PPL sera d'ailleurs poursuivi lors d'une mission d'information sur la situation des secrétaires de mairie. Pour laquelle j'aurai le plaisir d'être rapporteur aux côtés de mes collègues, Catherine Di Folco, rapporteur de ce texte et Jérôme Durain. Et présidée par. lancé par la délégation à l'aux collectivités territoriales la décentralisation présidée par Madame, Françoise Gatel, que je remercie aussi de son soutien. Cette mission a débuté ce matin lors d'une première, tables rondes et notre objectif sera de publier un rapport au cours de cet été où nous espérons dresser les recommandations à mener tant sur le plan législatif que réglementaires pour répondre au désarroi dans les territoires et embrasser le sujet dans toutes ses dimensions. Nous devons apporter des solutions concrètes tant pour répondre aux conditions de travail des secrétaires de mairie mais aussi pour rendre plus attractif ce métier tout en garantissant la continuité et de la visibilité, pour les mères. En effet, nous ne pourrons pas parler de statut de secrétaire de mairie sans aborder la formation initiale et continue, sans évoquer l'accompagnement notre secrétaire de mairie vers formations, qui doivent être concrètes et tourné vers la pratique du quotidien.

Là par les maintenant Madame, Colette Mélot pour le groupe les indépendants pour cinq minutes. Monsieur le président. Monsieur le Ministre, monsieur le président de la commission des lois. Madame la rapporteure. Mes chers collègues. L'urgent et fait l'impossible est en cours pour les miracles prévoir un délai ce panneau affichés dans la mairie d'une commune rurale reflète bien le quotidien d'une secrétaire de mairie. Les secrétaires de mairie sont les interlocutrice privilégiée de la population et vous me permettrez l'emploi du féminin. Puisqu'il s'agit pour l'immense majorité des femmes, de femmes. Ajoutons que le tandem que forment. Le ou la mère et sa secrétaire de mairie. Est un élément déterminant de la réussite du mandat municipal. Et nous avons la le 1er maillon de la République de proximité assurant le maintien du service public dans tous les territoires. Les secrétaires de mairie organise et assure l'accueil des usagers du service public et de nos administrés à réaliser les démarches administratives les plus essentielles, elles font le lien entre les citoyens et les élus. Je salue leur engagement quotidien et je remercie le groupe CRC. CRC d'avoir proposé cette. PPL disponible, accessible, elle participe à endiguer la fracture numérique. C'est tout particulièrement. Le cas en milieu rural où elle représente bien souvent l'unique guichet de proximité. Les secrétaires de mairie sont essentiels au bon fonctionnement des services publics locaux. Nous tous ici présents pouvons en témoigner pour en avoir côtoyé au cours de nos mandats et engagement dans nos territoires. Leur mission quotidiennes sont multiples, à l'image de la grande diversité de leur profil, la comptabilité, le montage des dossiers de de demandes de subventions. La réponse aux sollicitations diverses des habitants ou encore la gestion du personnel. Le parcours de formation dont bénéficient à ce jour les secrétaires de mairie est insuffisant sur le fond et inadapté. Sur la forme. Le Sénat, chambre des territoires s'est fait l'écho des remontées des associations d'élus locaux. Si je salue l'initiative du dépôt de cette proposition de loi, force est de constater que le texte initial souffrait d'un certain nombre de lacunes. Les amendements de la rapporteure dont je salue le travail. Pallier les failles évoqué. En commission. Le texte que nous examinons aujourd'hui apporte de vraies améliorations à l'exercice de ce métier de plus en plus complexes. La création d'une formation obligatoire est une avancée concrète, elle sera dispensée à l'ensemble des secrétaires de mairie de France par le Centre national de la fonction publique territoriale. Nous pouvons nous en féliciter. Méconnu parfois délaissée elles sont le coeur battant de nos communes. Notamment les plus petites d'entre elles. Il est donc essentiel d'apporter des réponses au manque d'attractivité de leur poste aux difficultés de recrutement et à la pénibilité de l'exercice de leur mission. Accompagner face à la digitalisation des démarches administratives actualiser les compétences développer de nouveaux savoirs échanger sur les bonnes pratiques. Autant d'objectifs auxquels les évolutions permise par ce texte permettront d'apporter des réponses pour ces raisons le groupe les indépendants votera favorablement cette proposition de loi modifié en commission. Ça ne vous en remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à monsieur Guy Bénard Roche pour le groupe écologiste pour cinq minutes. minutes. Le président. Monsieur le Ministre, Mesdames, messieurs les auteurs madame la rapporteure, chers collègues. À l'heure où le fait politique n'est plus compris et où l'élue de proximité de beurre l'élu préféré des Français. L'action concrète du maire au plus proche du quotidien de nos concitoyens l'écoute permanente. Auprès des administrés État Délia les plus solides qui perdure, alors que beaucoup trop de Français sont perdus dans le, comment ça marche d'un mille-feuille territorial dont ils se demandent le fonctionnement et parfois la légitimité. Le PPL qui nous est proposé de débattre aujourd'hui porte sur un des rouages clés du fonctionnement de cet échelon local si essentielle pour les petites communes. Le poste de secrétaire de mairie. Véritable outil d'interface entre les élus et l'administration et les citoyens. Ce poste remplis par des femmes en très grande majorité 94% de bénéficie pas de cadre ou statut à hauteur des missions qui lui sont dévolus. Ce manque de reconnaissance pourraient accroître les difficultés de recrutement dans les prochaines années vu l'âge moyen de 50 ans aujourd'hui de ce personnel qui existe déjà d'ailleurs au vu des près de 2000 postes vacants. Nos collègues du groupe communiste ont tenté d'apporter une solution à ce problème latent en proposant un statut innovantes pour ses employés essentiel au bon fonctionnement de l'autre territoire particulièrement comme le rappeler la rapporteure au fonctionnement des communes de moins de 2000 habitants qui représentent plus de 3 quarts des communes françaises. Les travaux de la commission ont modifié le texte mais l'urgence d'agir en faveur de la revalorisation de ses fonctions, hé bien là je regrette quelque part le refus de la commission de créer un statut spécifique mais je remercie notre rapporteur qui a fait état lors de ses travaux en commission ayant mené à la suppression des 3 premiers articles que je vous cite les dispositions relatives aux cadres d'intitulé conditions d'accès gris. Indiciaires ne relève toutefois pas de la compétence du législateur et a donc préféré substituer au dispositif proposé l'instauration d'une formation initiale commune à l'ensemble des secrétaires de mairie, quel que soit leur statut, ainsi qu'une mesure visant à favoriser la promotion interne des agents exerçant ses fonctions. Le choix d'étendre aux communes de 1000 à 2000 habitants. La possibilité de recruter sous forme contractuelle pour ces employes me semble toutefois un aménagement insuffisant. Le temps des mesures ponctuelles doit se terminer nous ferons appel au gouvernement, à cet effet et remplacée par une reconnaissance spécifique de ce poste-là contrat le la grande échelle, nous a toujours posé des problèmes vous le savez. Étant donné que les 2 tiers de ses personnels exercent à temps partiel et que près Dakar travaille sur plusieurs communes, nous aurions préféré. Une réflexion. Plus étendue et nous comptons encore une fois sur Monsieur le Ministre, s'ils m'écoutent. Sur une mutualisation éventuelle au niveau inter-communautaires pour partager le personnel entre les communes. L'autre commission la râpée. Ce poste est exercée outre par des agents contractuels, par des fonctionnaires territoriaux appartenant à l'un des 4 Cadre d'emplois suivant, celui de secrétaire de Marie. Catégorie a mis en extinction 2021 celui des attachés territoriaux catégorie à celui des rédacteurs territoriaux catégorie B et celui des adjoints administratifs catégorie C pour autant. Nous partageons avec tous le constat et la volonté de sécuriser au mieux le fonctionnement des mairies vers la pérennisation et la valorisation des secrétaires de mairie la pérennisation la visibilité dans les perspectives de carrière et de formation de ces postes particuliers sur la clé de consolidation et de la reconnaissance de leur travail. La spécificité du rôle de secrétaire de mairie nécessite une formation que notre commission a choisi à juste titre de généraliser et ce quel que soit le cadre d'emploi formation dispensée par le ciel FPT, le Centre national de la fonction publique territoriale. Je profite du temps de cette discussion générale pour saluer le dévouement de ces personnels véritable clé de voûte de l'échelon local dont l'appui juridique, administratif et technique particulièrement lors de la préparation des Budgets permette le bon fonctionnement de nos communes et leurs actions et politique locale, notre groupe votera donc ce texte et à son tour appelle le gouvernement à se saisir enfin pleinement et rapidement de ces questions majeures d'agents à qui nous devrions permettent plus que jamais de travailler dans des conditions dignes et convenables afin d'assurer un service public de qualité et accessible pour tous. Tout comme la commission nous encourageons donc le gouvernement a bien prendre en compte les rémunérations et parcours professionnel de ces personnes dans le cadre des travaux portant sur l'accès, la rémunération et les parcours professionnels dans la fonction publique lancé le 1er février dernier par le ministère de la transformation et de la fonction publique. Merci, cher collègue, la parole est maintenant au président Alain Richard pour le groupe RDPI pour six minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Indispensable. C'est un terme que nous utilisons dans bien des circonstances et parfois de façon un peu imagé. Mais dans le cas du Cadre d'emploi ou de la fonction territoriale dont nous parlons, le terme est vraiment à prendre au sens propre, on ne peut pas se dispenser. Des secrétaires de mairie de ses agents polyvalents qui assure le support administratif. Et légal de toutes nos collectivités. Il me semble donc c'est très heureux que nous ayons. À partir de la proposition de loi de nos collègues communistes. Un débat sur ce sur tout ce que nous envisagions la vraie conclusion de ce débat et. Comme d'autres collègues je sais bien que cette conclusion elle nous met en relation directe avec le gouvernement. La première chose sur laquelle il faut je crois progressé c'est une. Et d'ailleurs le ministre l'a dit tout à l'heure une redéfinition de l'emploi. Il faut mieux caractériser et actualiser l'ensemble des aptitudes et l'ensemble des fonctions que recouvre cet emploi de manière que. Le profil et le support de recrutement soient claires pour l'avenir ils tiennent compte de de toutes les transformations que nous avons. Vu et opéré d'ailleurs. Mais. Nous sommes à un moment où nous voyons les limites de la de la l'édifice statutaire. Le système statutaire et d'abord une garantie de droits professionnel il est assorti d'un schéma. Conçu par nos anciens. À la Libération fondé sur une nomenclature de l'intégralité. Des emplois et des grades assortie d'une échelle indiciaire qui est. Complètement uniformes. Nous voyons bien et je ne sais pas d'hier. Au cours de ma carrière administrative. Je l'ai vu dans 50 circonstances. Depuis que sont apparus des spécialités ou des. des. Spécificités professionnelles qui échappaient à ce à cette grille initiale. Il y a qu'une solution, on le sait tous, elle s'appelle la contractualisation. Et donc. Il faut bien entendu que nous fassions le maximum pour rétablir une attractivité et une visibilité durable de ses fonctions. Donc il faut commencer par assurer que la totalité des personnes qui exercent en tout cas de manière permanente. Et professionnelle cette fonction sortent de la catégorie C, ça n'a plus aucun sens. Le niveau de qualification requis. Hé bien au-dessus de ce que représente la catégorie C, donc il faudra faire fonctionner il faut l'organiser de façon urgente un schéma de reclassement fondée sur la reconnaissance des acquis. De l'expérience pour l'ensemble de ses personnels. Il faut ensuite que nous fassions du hors norme. En ce qui concerne la rémunération puisque nous voyons bien. Que les marges du Rif ne sont pas suffisantes et ne permettront pas, compte tenu des différents systèmes de chaînage des indices. Qui l'encadrent. Nous savons bien que nous n'arriverons pas au niveau de d'attractivité de de comment dire de, de reconnaissance de la fonction suffisante et puis donc nous serons amenés sans doute et c'est un des points positifs de cette proposition de loi, de dire que on peut recruter sur contrat. Et donc avec une marge et de d'appréciation sur la rémunération. La. L'ensemble des personnels, secrétaire de mairie jusqu'à 2000 habitants. Je voudrais ajouter une composante qui est peut-être. Plus perçu perceptible dans la périphérie dans les zones périphériques des grandes villes où il y a une tension immobilière importante. Le droit actuel, Monsieur le Ministre ne permet pas à une commune de loger sa secrétaire de mairie. Je remercie d'ailleurs le rapporteur de m'avoir. Donné un coup de main pour clarifier ce droit. Une une mairie qui loge. Sa secrétaire de mairie ou qui d'ailleurs lui c'est une, un contrat de location avec un loyer très inférieur au prix du marché comme une illégalité. Et donc il faut certainement, puisque ce sera un élément de l'attractivité de la, de la possibilité réelle d'exercer cet emploi dans le cours d'une carrière. Il faut certainement que vous libérer aussi ce Je pense donc. Il va y avoir des conséquences sur les finances communales selon nous parlons. Et donc. Monsieur le Ministre. Je crois qu'on peut vous donner rendez-vous. À la prochaine loi de finances. Il faut que le, le paquet de mesures. Destinées à rétablir l'attractivité et la visibilité de ses fonctions soit bouclé. Avant l'été. Et que comme il y aura des conséquences, j'imagine. J'imagine. Que 30.000 communes. Et en moyenne. Un surcoût lié à ces mesures. De 2 ou 3000 euros annuels. Qui s'étale par exemple entre les années 2024 et 2025. Il me paraîtrait légitime que ceux-ci fassent l'objet d'un chapitre dans une catégorie au sein du calcul de la DGF, c'est pour ça, il me semble judicieux de vous donner rendez-vous avant la loi de finances, merci. Merci. Le ministre a pris rendez-vous naturellement. Et la parole est à monsieur Hussein Bourgi pour le groupe socialiste pour cinq minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la rapporteure. Monsieur le président de la commission des lois, chers collègues. Se salit notre collègue Céline Brulin, et ses camarades du groupe CRCE pour cette initiative qui nous permet aujourd'hui de répondre à quelques-unes des attentes de secrétaire de mairie qui est qui officie dans nos communes. Je veux saluer aussi Catherine Di Folco, rapporteur de la commission des lois pour l'exhaustivité et la richesse des auditions qu'elle a mené. Cette proposition de loi est particulièrement bienvenue car elle nous donne l'occasion de nous pencher sur le sort de secrétaire de mairie ce métier méconnu. Oh, peu connu du grand public mais ô combien précieux dans les communes. En effet, que serait une équipe municipale son secrétaire de mairie. À la fois juristes fiscalistes trésorier et trésorière urbaniste rédacteurs et rédactrices mais aussi parfois assistantes sociales, psychologues, conseillers et conseillères d'orientation. Le secrétaire de mairie représente bien souvent dans nos communes. L'incarnation du service public municipal, un service public à visage humain. Accessible à toutes et à tous. Le secrétaire de mairie et souvent dans les villages appeler par son prénom. C'est dire le lien si fort qui unit la population au secrétaire de mairie. Le secrétaire de mairie sont aussi au quotidien les partenaires du maire et de l'équipe municipale c'est personnels, aide à la conception et à la mise en oeuvre des décisions des élus. Le secrétaire de mairie contribue donc à l'efficience des politiques publiques locales aussi, disons-le sans flagornerie et sans ambages, sans le secrétaire de mairie les communes notamment dans le milieu rural n'existerait simplement plus. Pourtant malgré son intérêt et sa polyvalence ce métier qu'on connaît une perte d'attractivité évidente, si bien que les collectivités notamment celles de moins de 2000 peinent à recruter. Que dire de celles de moins de 1000. Les perspectives sont inquiétantes. D'ici 2030, un quart de secrétaire de mairie partira à la retraite et pas de renouvellement générationnel assuré à ce jour. Alors je vous le dis, mes chers collègues, je vous le dis, Monsieur le Ministre, si on rajoute la crise de vocation chez le secrétaire de mairie à la crise de vocation chez les élus et chez les maires en particulier on va droit à la catastrophe. Venons-en 3 articles qui reste. Soumis à notre. Travail aujourd'hui à notre examen. L'article 4 prévoit une formation obligatoire dispensée par le Cnfpt pour l'ensemble des secrétaires de mairie, dans un délai d'un an. À compter de leur prise de poste. Cet article confère un caractère indispensable. Information il est bienvenu au regard de la multiplicité des tâches que devront accomplir ses personnels et au regard de la complexification permanente de la législation et de la réglementation. Pour autant, le dispositif voté en commission n'évoque pas le régime d'absence qui encadrerait son application. Il va sans dire que ce silence pourrait mettre à mal l'efficience de cette mesure. L'article 5 vise à garantir des perspectives d'évolution de carrière pour cette profession. En prévoyant une part de secrétaire de mairie sur l'établissement des listes d'aptitudes. C'est un des leviers pour favoriser l'évolution de carrière de secrétaire de mairie et il est donc bienvenue. Enfin, nous sommes plus réservés quant à la philosophie de l'article 5 bis. Si nous comprenons et connaissant les difficultés de recrutement dans les communes de moins de 2000 habitants, nous ne sommes pas pour autant convaincu de l'utilité de permettre le recrutement de contractuels dans ces communes-là. Relèvement du plafond des communes de moins de 1000 à moins de 2000 reviendrait tout simplement à répartir la pénurie et conduirait à une forme de concurrence entre les communes de 1000 à 2000 habitants qui ont parfois quelques moyens un peu plus important que les communes de moins de 1000 habitants. Au groupe socialiste, écologiste et républicain. Nous restons persuadés que d'autres moyens peuvent être envisagées pour redonner à la profession son attractivité le 1er levier, celui de la rémunération, un effort a été fait, Monsieur le Ministre, avec le décret du 28 février 2022 sur la NBI pour les postes de secrétaire de mairie au sein des communes de moins de 2000 habitants. Mais cette mesure se heurte à 2 écueils. Elle reste tout d'abord insuffisante pour atteindre un niveau de rémunération descend au regard des responsabilités ensuite la charge de cette revalorisation est porté par les collectivités locales qui n'ont souvent pas les moyens de financer une telle disposition est compris lorsque plusieurs communes. La même secrétaire de mairie dans mon département dans les roches et des secrétaires de mairie qui sont salariés par 3 ou 4 communes mais elles n'ont pas un temps plein et chacun se renvoie la balle pour appliquer cette nouvelle mesure. L'article 6 de cette proposition de loi apporter un début de réponse avec la création d'un fonds de soutien local la forme du dispositif mais qui est sans doute pas la bonne. La question soulevée aurait mérité un débat ici en séance. C'est la raison pour laquelle je pense que lors du PLF, et comme l'a dit le ministre Alain Richard. Nous aurons l'occasion d'y revenir, Monsieur le Ministre. Le sujet est trop sérieux, on ne peut pas se permettre d'avoir un jeu de ping-pong permanent entre vous monsieur Attal monsieur Béchu et Madame fort, il va falloir que le gouvernement s'accordent sur cette question pour qu'on réponde vraiment sérieusement et franchement à cette préoccupation majeure. Chez tous les élus municipaux concernés par ce problème, vous l'avez compris, Monsieur le Ministre, Mesdames, messieurs, chers collègues, nous voterons favorablement cette proposition de loi en prenant date pour l'avenir. Merci à tous et à toutes. Merci, cher collègue, la parole est maintenant au président Jean-François Longeot pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il est grand temps que nous prenions en compte l'importance du rôle stratégique que joue les secrétaires de mairie dans notre pays. Il m'est donc impossible de commencer sans saluer l'initiative de nos collègues du groupe CRCE. Qui contribue à mettre sur le devant de la scène. La situation de de secrétaire de mairie. C'est 14.000 agents publics souvent les femmes sont les gardiens des bases administrative de nos villages et de nos communes. Ils sont les premiers acteurs de notre société à être en contact Direct avec les citoyens. Ils reçoivent et traitent leur demande leurs réclamations leurs doléances. Ses secrétaires sont les collaboratrices directe du maire et de la municipalité. Elles oeuvrent au bon fonctionnement du service public local chaque jour sans compter ni leur temps, ni leurs heures et joue ce rôle si essentiel de trait d'union entre les administrés. Les élus et les autres administrations. Malheureusement ce métier n'est pas suffisamment reconnu. Les secrétaires de mairie sont souvent considérés comme des employés administrative excusez-moi du terme de bas niveau. Alors qu'en réalité elles sont, elles ont des responsabilités bien plus importante. Hé bien plus élargie. En effet, elles organisent des services de la commune. laveur concrètement le budget gère ses ressources humaines. L'état civil l'urbaniste les délibérations, les arrêter et cetera. De plus ces secrétaire municipal doivent constamment s'adapter à la complexité aux mutations des procédures administratives. Faute de candidature le recrutement de secrétaires de mairie s'avère de plus en plus difficile. Les causes je crois sont connus exigences techniques et juridiques d'. Rémunération trop faible. Obligation de cumuler plusieurs postes pour parvenir à un temps plein. Cette pénurie risque de s'aggraver car et ça a été dit. Un tiers des secrétaires de mairie en poste partiront à la retraite d'ici 2030. Il est donc temps de prendre des mesures concrètes pour revaloriser le statut des secrétaires de mairie en France. Nous devons reconnaître leur importance et leur rôle crucial dans l'administration locale en leur offrant une formation adaptée, une formation adéquate et en leur octroyant des primes et des augmentations de salaire à la hauteur de leurs compétences. De plus, nous devons également voir leur classification et leur faire bénéficier d'une progression de carrière qui prennent en compte l'ancienneté et les compétences acquises. Enfin, il est urgent de mettre en place des dispositifs de sécurité appropriées pour garantir leur sécurité au travail. Faire face aux incivilités ou aux agressions physiques dont elles peuvent être victimes de plus en plus fréquemment. Pour conclure je dirais qu'il nous faut rendre plus attractif ce métier mais qui est très diversifié qui demande de nombreuses qualités sur le plan professionnel, et sur le plan humain. Les secrétaires de mairie sont un maillon incontournable de la vie communale. Et sont l'avenir également de nos communes. Il devient plus qu'urgent de leur donner la reconnaissance qu'elle mérite. Ce serait là un investissement essentiel pour le bon fonctionnement de nos collectivités. Et comme l'a dit ma collègue Nathalie Goulet. Le groupe UC votera sans aucune. Hésitation en faveur de ce texte. Je vous remercie. La parole est maintenant madame Béatrice Gosselin pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Monsieur le président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Comme cela a déjà été rappelé le poste de secrétaire de mairie et c'est lui le plus en tension de la fonction publique territoriale. Alors que cette profession est indispensable au bon fonctionnement de l'administration de nos communes rurales, le métier souffre d'un manque de reconnaissance comme d'une profonde méconnaissance de la règle sur la réalité des fonctions exercées. Le secrétaire de mairie assurent des tâches essentielles en matière de budget d'état civil d'élections et de recensement de gestion funéraire ou encore d'urbanisme et de marchés publics. Et parfois il gère aussi les ressources humaines de la commune. Toutes ces tâches s'effectue évidemment en même temps que l'accueil du public. Véritable couteau suisse de nos collègues de nos petites collectivités, ce sont les premières personnes que l'administrer rencontrent lorsqu'il se heurte à une difficulté dans sa commune. Sur les 368 communes de moins de 2000 habitants de la Manche, 260 ont un seul agent et pour plus des 2 tiers. Ce sont des adjoints administratifs de catégorie C. De cette spécificité statutaire sans équivalent pour d'autres métiers de la fonction publique découle notamment l'absence de concours propre au métier de secrétaire de mairie et donc un certain manque de visibilité pour des candidats éventuels. Et sur le terrain nous le constatons les secrétaires de mairie sont dans leur quasi-totalité des femmes et relèvent majoritairement de la catégorie C. La plupart d'entre eux travaillent de manière isolée et son secrétaire à temps partiel de 2 ou 3 mairies différentes au cours de la semaine

D'ailleurs certains EPCI consciente du déficit d'attractivité, d'un emploi à temps partiel favorise les postes à temps complet en proposant une mutualisation des horaires. Sur plusieurs petites communes. Enfin l'appellation secrétaire de mairie apparaît aujourd'hui quelque peu désuète et ne correspond assurément plus à la nature des fonctions exercées par des agents concernés. Cependant ce titre évoque un sentiment d'accessibilité, de proximité et reste publicité par des habitants. Alors quelles sont les pistes envisageables pour remédier à ces problèmes d'attractivité, d'autant plus sensible dans un contexte de quasi plein emploi comme celui de la Manche. Plutôt que de créer un soutien à fond de soutien à. Comme le prévoyait à l'origine de la proposition de loi. La commission des lois, ouvert aux communes de moins de 2000 habitants la possibilité de recruter des contractuels pour leurs emplois permanents de secrétaire de mairie. Cette disposition n'était pas possible avant. N'était possible auparavant que pour les communes n'excédant pas 1000 habitants. Il est également plus pertinent de privilégier l'autonomie financière des communes qui ne doit pas passer par une compensation mais par une fiscalité adaptée, ainsi que l'indexation de la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation. S'il n'existe pas de concours propre au métier de secrétaire de mairie une formation académique consacrée à ce métier destiné aussi bien aux étudiants qu'à des actifs en reconversion professionnelle est en cours de développement. Certaines universités organisent en effet en partenariat avec les centres de gestion des formations en alternance qui conduisent à l'octroi d'un diplôme universitaire. C'est le cas avec la licence professionnelle métiers de l'administration, des collectivités territoriales du pôle universitaire Un partenariat entre Pôle emploi et le Cnfpt qui associerait également Association des maires de. France et l'association de régions de France pourrait permettre la mise en oeuvre de formation au métier de secrétaire de mairie à destination des membres demandeurs d'emploi. Toutes ces initiatives ou pistes envisageables ne saurait nous dispenser d'une réflexion de fond sur les moyens. Ah mais d'améliorer l'attractivité de la fonction publique territoriale. Les employeurs publics et notamment les employeurs territoriaux doivent avoir une véritable politique de communication pour mettre en avant l'extrême variété des métiers proposés et des carrières mener. Enfin et surtout les récentes mesures ponctuelles de revalorisation reste limitée dans les faits, seule une véritable réforme globale des règles de rémunération pourrait rendre cette profession plus attractive. S'agissant de la promotion interne. Le ministère le Ministre de la transformation et de la fonction publique a récemment indiqué que le projet de refonte des modalités d'accès de parcours et de rémunération intégrera une réflexion sur les règles de promotions dans la fonction publique territoriale à laquelle les employeurs territoriaux ressent. Et je m'en félicite. Ainsi il pourrait être proposé que des centres de gestion fixe les quotas selon les besoins locaux, en terme d'emplois. Enfin, l'État pourrait envisager des modalités d'accompagnement financier des centres de gestion qui s'engagent dans des initiatives innovantes comme en développant la mission de tutorat. Je voulais saluer l'excellent travail de nos collègues du CRCE et du rapporteur Madame Catherine Di Folco qui pose les bases de ce de ce métier c'est la réforme de ce métier est une. Permettra une revalorisation essentiel et cette refonte j'espère sera à la hauteur des espérances que ce que voudrait la profession le groupe des Républicains votera le texte modifié par l'Europe. Le rapporteur, je vous remercie. Merci cher collègue. Là. Par les maintenant monsieur Rémy Cardon. Pour le groupe socialiste pour 4 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues. Je souhaite débuter cette intervention en rendant justement hommage à notre collègue et Céline Brulin, et à ses collègues également ses camarades du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Qui ont fait d'ailleurs le choix de d'utiliser leur niche parlementaire pour mettre en lumière cette profession qui a une réelle importance dans nos territoires. En effet la réalité du poste de secrétaire de mairie hé bien plus vaste que nous serions imaginer le elle parce que la profession est à 94% féminine. N'auront plus ce lien précieux qui unit au quotidien citoyen et République. Hier. Elles étaient les couteaux suisses de la République, elles le sont toujours. Mais aujourd'hui, elles sont devenues les perles rares de la République. À la fois par leurs compétences de juriste trésorière urbanistes ou encore rédactrice et surtout. D'assistante sociale, parfois pour des cas exceptionnels ou encore. Conseillère numérique puisque elle joue aussi un rôle. Au plus près dans certaines communes quand il y a un manque de de France services ou de ou de service public. En tout cas, ce sont à la fois le 1er et le dernier visage du service public municipal accessible à tous nos concitoyens. Au quotidien elle mènent un travail et en texte et elles permettent à nos villes à nos villages de vivre sur en tant que entité politique et administrative fonctionnelles elles apportent un appui technique et humain précieux qui participent à la vie de nos communes et qui donne pleinement. Du sens à la promesse républicaine. Et pourtant ce maillon essentiel. Du lien entre la République et les citoyens n'est pas valorisée à sa juste valeur. Faible rémunération statuts précaires. Multiplication des temps partiels et des difficultés attacher ce métier connaît une perte d'attractivité évidente, si bien que les collectivités, notamment celle de notamment de moins de 1000 habitants peinent à recruter. Elle manquerait aujourd'hui effectivement près de. 1009 1900. Secrétaire de mes mérites dans tout le territoire et d'ici 2030. Vous l'avez, vous l'avez dit, chers collègues, ce sont plus d'un tiers des secrétaires de mairie qui partiront à la retraite sans qui un renouvellement générationnel assumer au sein de la profession. Alors cette proposition de loi entend poser le 1er jalon d'une revalorisation du statut de secrétaire de mairie et nous accueillons positivement. Et même si le sujet de la revalorisation des secrétaires de mairie ne relève quasi exclusivement du domaine réglementaire, cette proposition ouvre au moins un débat utile sur l'attractivité de ce métier décisive pour nos collectivités est essentiel pour notre République. Nous pourrons donc attends. En tout cas des amendements adoptés en commission des lois. Madame la rapporteur a. Pris soin de de donner quelques apports en tout cas, de le rendre le texte plus opérationnel. Nous l'avons compris même si effectivement on peut perdre un peu de sens en la matière. Je vais pas revenir sur. Le différend. Faire un focus sur les différents contenus puisque mon cher mon collègue et c'est une Bourget en a fait une. Grosse part en tout cas, nous pensons que, avec le groupe socialiste, écologiste et républicain. Que d'autres pistes permettent de valoriser. Cette profession. Elles devront être étudiées. Ça peut commencer par un premier levier que vous avez cité. Les uns après les autres la rémunération. Bien qu'il ait eu effectivement un effort, par le biais du décret. Donc le 28 février 2022, juste avant les présidentielles. Cela reste très voire trop insuffisant. Cette mesure d'ailleurs, se heurte en réalité à 2 écueils. La première effectivement une augmentation de 70% brut par mois armée-nation n'atteint toujours pas le niveau décent au regard des responsabilités porté au au quotidien par par celle-ci. Et ensuite la charge de cette revalorisation est portée et ça a été dit par les collectivités locales et donc je soulève la proposition de monsieur. Alain Richard, sur le fait qu'il va falloir regarder ça de près sur le PLS également. À ce sujet le gouvernement peut et doit. Et c'est mieux faire mais c'est terminé. Allez je vous remercie. La parole est maintenant Madame Véronique Del Fabbro pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes.

Monsieur le président. Monsieur le Ministre. Monsieur le président de commission, madame le rapporteur, mes chers collègues. Le constat est alarmant d'ici 2026, date du début du prochain mandat municipal, ce sont plus de 150, secrétaire de mairie en poste dans des communes de Meurthe et Moselle qui partiront à la retraite. 80% des communes de ce département possède moins de 2000 habitants. Mais il n'est pas une exception car, à l'échelon national, ce sont 42% des secrétaires de mairie qui partiront dans les 10 prochaines années, le métier de secrétaire de mairie peu valoriser et complexe sous d'attractivité comme on l'a entendu précédemment et les mairies font face aujourd'hui à une pénurie sont disposées vraiment de moyens pour y remédier le secrétaire ou plutôt la secrétaire est un collaborateur Direct et et son ciel du maire, c'est véritablement un relais pour les habitants. Elles sont le savoir des communes et bien souvent la mémoire. Les élus passent les secrétaires reste l'accroissement des compétences communales et intercommunales fait considérablement évoluer ce métier les tâches effectuées à ce poste sont diverses et variées et dans l'élaboration du budget, suivi du budget, gestions des ressources humaines, rédaction du courrier. Civilistes. Électorale cimetière. Je vais arrêter là, mais vous avez bien compris certaines même des secrétaires de mairie montent les dossiers de subvention et même des dossiers de subvention fédère. bien qu'indispensable. Ces professionnels ne sont pas suffisamment connus et reconnus à leur juste valeur les raisons de cette pénurie sont nombreuses et mes chers collègues, vous les avez déjà évoqué comme le manque d'attractivité du métier, la faible rémunération, le temps partiel nous que nos chers secrétaire de mairie occupent des postes dans des petites communes dans des syndicats doivent travailler sur des outils différents, avec des préfectures différentes des intercommunalités différentes des trésoreries différents ce qui nécessite de leur part une très grande adaptabilité. N'oublions pas le mal-être qui est palpable. Les réseaux sociaux valent ce qu'ils sont. Je suis d'accord mais ils sont révélateurs d'un malaise et d'un mal-être lorsque l'on lit leurs posts sur le groupe Facebook que certaines anime. Changer l'intitulé du poste n'est pas la solution. Monsieur le Ministre mais c'est une solution pour refléter davantage la réalité et les responsabilités de ce métier. Un autre aspect combien important et la formation, l'information initiale en Meurthe-et-Moselle, centre de gestion a décidé de créer en 2018 en partenariat avec l'Université de Lorraine, un diplôme universitaire intitulé secrétaire de mairie, gestionnaire administratif. y ait une formation Californie qualifiant pardon diplômante qui permet d'apporter des connaissances. Théoriques et pratiques puisque le stage de huit mois et bien souvent effectués dans la commune pour laquelle la secrétaire de mairie va partir en retraite. Le taux d'insertion professionnelle et de 90%, il est nécessaire de dupliquer ce diplôme universitaire et mon choix au niveau national pour tenter de répondre à la pénurie de la profession. Les moyens des communes rurales étant limitée et pour lutter contre cette précarité, certaines communes n'hésite pas à mutualiser le recrutement afin d'offrir à ces femmes des postes à temps complet davantage des avantages sociaux et même une formation. Cette formation est un enjeu pour la bonne continuité du service public, ce qui est d'autant plus vrai pour les petites mairies, nous devons offrir à ces personnels, des conditions de travail décentes des rémunérations juste des formations régulières pour le permettre de s'adapter aux évolutions du métier. Cela permettra de garantir un service public de qualité et d'assurer la continuité de nos communes. C'est pourquoi le groupe Les Républicains est favorable à ces 2 propositions de loi et remercie le groupe communiste de l'avoir proposé telle qu'elle a été modifiée par la commission. Merci. Merci. La discussion générale est Close. Je passe au texte de la commission. L'article 1er supprimé l'article 2 de supprimer l'article 3 est supprimé à l'article IV. J'ai plusieurs demandes de prise de parole madame la présidente Françoise Gatel d'abord. Merci monsieur le président, monsieur le ministre. Monsieur le président, madame la rapporteure et suis vraiment saluer l'initiative de notre collègue Céline Brulin, et de du groupe CRCE, c'est une proposition bienvenue parce qu'elle met sous les projecteurs. Cette fonction de secrétaire de mairie qui constituent chacun lundi un maillon essentiel de l'action publique de proximité en difficulté ce qui participe certainement à la fatigue des mères cette PPL. Nourrira sans aucun doute le travail qui vient d'être lancée ce matin par la délégation aux collectivités territoriales et qui sera conduit par Catherine Di Folco, Jérôme Durain et Cédric Vial sur l'attractivité de la fonction territoriale attirer et fidéliser voilà 2 défis nouveau pour nos collectivités. Et les candidats ont de préoccupations Jérôme Durain les expliquer d'une manière très claire en 2 mots, c'est le sens du travail mais aussi les sous-, c'est-à-dire la rémunération et face à ces difficultés. Je crois qu'il convient de chasser en meute et d'éviter de se concurrencer entre types de collectivités. C'est pourquoi je voudrais saluer les initiatives qui ont été prises par certains territoires. Alors Monsieur le Président. À tout seigneur tout honneur, je parlerai d'abord de vous il y a une marque de territoire qui a été créé, qui s'appelle Only Lyon une marque de territoire aussi qui a été créé en Bretagne. Pardonnez-moi, qui s'appelle Le den BZH comme tout le monde le sait, tout le monde parle le breton. Je vous donnerai le sens des choses après c'est une marque de territoire qui permet à 400 de gestion de se regrouper aujourd'hui cela concerne 2200 collectivités. Plus de 9000 agents s'est développé de l'attractivité du savoir-faire à l'échelle d'un territoire. Je vous remercie. Mais merci, la parole est à monsieur Philippe Folliot. Merci monsieur le président. Monsieur le Ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord saluer notre collègue Cécile Céline pour son initiative parce que c'est une initiative particulièrement importante et qui correspond à des besoins qu'ils ont des besoins éminemment n'a exprimé par d'une part les secrétaires de mairie elles-mêmes mais aussi il faut le dire par les mères parce que. Dans les communes rurales pour que ça fonctionne bien. Si vous me permettez, c'est le duo secrétaire de mairie mère et qui fait que les choses se passent et fonctionne bien. Dans le cadre de ce texte et et je prends. Prenant acte du fait que la commission et décidé de supprimer les articles 2 et 3 mai au travers de ses articles 1 2 et 3. Je crois que l'auteur de la proposition de loi poser de vraies questions et qu'il nous appartiendra collectivement d'essayer de trouver des solutions pour faire de telle sorte notamment par rapport au avoir un cadre spécifique adapté donc pour les secrétaires de mairie, que l'on puisse trouver les solutions on se félicite du travail qui va être menée, notamment au sein de la délégation aux. Territoriales donc aux collectivités territoriales de notre assemblée. Pour autant, cet article pose la question de la formation et c'est un élément qui est un élément essentiel. Mais moi je voudrais attirer votre attention sur un point et un élément de spécificités notamment dans les communes qui ont. Un seul agent qui est secrétaire de mairie. Ce droit à la formation et cette nécessité qu'on va inscrire donc dans la loi, il faudrait qu'il puisse être effectif et pour qui sur effectif il y a un enjeu et un élément, c'est que quand vous avez un seul agent si cet agent va. Ça veut dire de fait de fermer la mairie, et donc se pose la question du remplacement donc de de l'agent. De la secrétaire de mairie qui va faire valoir ce droit à la formation. J'avais déposé un amendement qui je regrette ben on n'a pas pu être. Repris dans le cadre de l'article 40. Mais en tout état de cause, il va falloir que nous réfléchissions collectivement sur les solutions à apporter pour faire de telles sont. Ce droit à la formation soit effectif au travers de remplacement des agents. Merci c'est terminé.

excellent texte je je le dis. Et on inscrit dans le dans le marbre de la loi. La formation initiale notamment cette indispensable au regard de la multiplicité des tâches. Ça a été dit de la polyvalence que cela demande et puis de la complexité croissante effectivement. de ses missions. Cet article est d'autant plus important et nécessaire. Quand on regarde la situation actuelle en matière de formation. Je m'en entretenais il y a peu avec Jean-Pierre Gérardin le le président du Centre de gestion dans

quinzaine. Au regard. Hé bien des financements octroyés alors. En Bourgogne Franche-Comté, la région a a déployé des crédits pour permettre ces formations et et donc on voit bien, Le nombre de candidatures non satisfaite pour pouvoir suivre ces formations donc cet article 4 est un est un bon article, de ce point de vue là je pense qu'on n'échappera pas un débat également sur le financement, puisque vous l'avez vu. Cette là un financement volontaire de la région qui qui permet cela. Et je crois qu'il faut travailler. À des règles à une gouvernance pour le financement de ces actions de formation. Afin qu'elle soit véritablement. Mis en oeuvre et. Nul doute que ce sera. Un des sujets sur lesquels la mission d'information se penchera, je le dis puisque Cédric Vial être avec nous dans, dans l'hémicycle. Et puis peut être un sujet de rendez-vous effectivement dans la loi de finances, je vous remercie monsieur le président. Merci cher collègue. 2 amendements en discussion commune le hein Madame Goulet. Oui, monsieur le président, Monsieur mais j'avais évoqué ça pendant la discussion générale, saisie d'un amendement d'appel sur le nom des secrétaires de mairie. Alors moi il va souffler par le président du Centre de gestion de l'iode mais de l'ordre. qui considère qu'il s'agit plutôt de collaborateurs communaux. C'est un amendement d'appel qui vaut ce qu'il vaut, qui sera probablement retiré puisqu'on a discuté déjà du sujet, tout à l'heure mais il est quand même il est quand même soutenu. Monsieur le président, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues. Pourquoi consacrer autant de temps. Dans le débat. À parler du titre et de la fonction de secrétaire de mairie, tout simplement, c'est une demande des personnels concernés. Le titre la fonction c'est la carte d'identité professionnelle, c'est la carte de visite de ces hommes et de ces femmes. Il se trouve que je suis délégué du Cnfpt en région Occitanie et depuis 3 ans, je suis amené à accompagner dans le cadre de la convention et du partenariat que vous avez appelé de vos voeux Monsieur le Ministre entre le Cnfpt Pôle emploi. Le Centre de gestion et l'Association des maires. J'ai été amené à accompagner, à peu près 500 personnes. Et lorsqu'on fait les le questionnaire de d'évaluation et de satisfaction à la fin de la formation. On pose la question du nom. Alors lorsque vous leur parlez de collaborateurs de collaboratrices du maire ils disent ça a une connotation une coloration politique lorsque vous leur parlez de secrétaire de mairie, vous dites je ne suis pas la secrétaire ou le secrétaire du maire. DGS le DGS des grandes collectivités ne veulent pas en entendre parler. Ça peut s'entendre et se comprendre. Responsable du personnel communal, les maires ne veulent pas entendre parler parce que ce sont les maires, les responsables du personnel communal et donc le seul titre la seule fonction qui fait consensus sur ce panel de 500 personnes qui aspirent à exercer ses fonctions. Mais j'ai pu le corréler aussi avec le secrétaire de mairie qui sont elles et eux actuellement en poste lorsqu'il vient se faire former. Dans le cas de la formation continue sur le 13 départements de la région Occitanie et je peux vous dire Monsieur le Ministre que je tiens à votre disposition les résultats de cette enquête et la proposition que je porte ici découle de ce questionnaire de satisfaction et de ce choix préférentiel qui ont été faits par le secrétaire de mairie. Merci. Avis de la commission, madame la rapporteure sur ces deux amendements. Merci, monsieur le Président, alors effectivement c'est un sujet hein. Cette appellation et et je comprends tout à fait l'intention des des auteurs mais c'est vrai que si l'appellation secrétaire de mairie paraît un peu Je l'ai entendu lors de la discussion générale qu'il ne correspond pas tout à fait maintenant aux aux missions qui sont exercées parce qu'elles vont au-delà du, du secrétariat. Sans doute faut-il un terme plus moderne. Vous avez, vous

l'assentiment général et en tout cas quand on a interrogé. Le, le syndicat des secrétaires de mairie. Elles-mêmes les anciennes secrétaires de mairie qui sont là depuis plus de 30 ans elles disent non c'est notre métier quoi on est attaché à notre métier. Ils n'ont pas forcément envie de le changer d'appellation. Donc c'est un peu complexe donc je propose que pour l'instant on on en reste là je j'émettrai un avis soit de retrait soit défavorable et retravailleront le sujet avec les intéressés, en particulier, je vous remercie.

Sans rien. De l'importance du changement de nom et la qualification du métier, je partage ce que vous avez dit monsieur sénateur c'est la carte de visite, c'est très important, mais en méthode je crois que c'est avec les secrétaires de mairie avec les associations d'élus, avec les employeurs territoriaux qu'on doit pouvoir définir le titre de ce métier là donc je serai aussi sur un avis. De retrait ou dans ce cas-là défavorable sur les différents types qui ont été proposées. Je pense que celui de. De de collaborateurs communal me semble un peu générique et pas forcément recouvrir de la diversité des fonctions et notamment celle de relations publiques. Qui convient ou qui conviendrait à ce métier de secrétaire de mairie d'autres intitulé existe dans le Champ des des propositions responsable administratif, secrétaire général de mairie mais ça doit être mis au débat, je pense qu'il a des idées qui peuvent être intéressantes dans ces 2 titres que je viens d'évoquer, mais je crois vraiment comme méthode, c'est avec les secrétaires de mairie que nous devrons décider donc avis. Aux demandes de retrait ou avis défavorable. Merci. Je vois qu'il y a plusieurs demandes de paroles. Je vais d'abord vérifier que les amendements ne soit pas. Madame Goulet. Première tirer le le l'amendement numéro 2 et retiré également. Merci. Monsieur. Il est maintenu, donc je donne la parole d'abord d'abord Madame brûle hein puis au président Alain Richard. Merci Merci monsieur le président. Je remercie les collègues qui par ces amendements. Contribue à la réflexion. Sur la dénomination l'appellation qu'on doit donner à ce métier de secrétaire de mairie. Nous nous y étions nous-mêmes essayer à travers le travail sur cette proposition de loi et pour tout vous dire ce que nous y a vu, on a même proposé ne nous semblait pas complètement satisfaisant. Donc moi j'entends ce que vous venez de dire monsieur le Ministre, comme un engagement de votre part à ce que des concertations soient menées avec les principales intéressées, évidemment avec les élus locaux et leurs associations pour qu'on parvienne à un nom qui disent mieux. Ce qu'est leur véritable fonction dans toute la polyvalence et toutes les responsabilités qu'on a évoqué depuis le début de cette discussion. Je nous met en garde collectivement qu'il ne faudrait pas que ce changement de nom. Combien même nous trouverions le nom parfait soit l'arbre qui cache la forêt. Parce que il y a d'énormes attentes. Et vous l'avez rappelé, les uns et les autres, notamment en terme de rémunération. Et je pense que changer de nom sans toucher à un iota. De la rémunération, ce serait mettre en colère les secrétaires mairie je vous le dis comme je le pense et donc dans l'engagement du travail de la réflexion autour de ce changement de nom, je pense qu'il faut y associer. La réflexion sur la rémunération qui me semble déterminante. Merci. Le président Richard. Mais je voudrais simplement signaler l'expérience que nous avons eue avec le changement du nom et du titre d'instituteurs. Surtout les vieux. Nous entend boules beaucoup de gens. Là le changement des nominations doit dater de 20 25 ans à peu près hein. Il y a encore une partie importante de la population qui continue à lire, instituteur. Donc quand on aura fait le changement ça s'appliquera de façon assez progressive. Madame la présidente Gatel. Monsieur le président. Alors je j'entends et je comprends et je partage nécessité sans doute de changer le mot. Qui a une connotation qui correspond plus vraiment au métier. Mais je rejoins ce que dit c'est une brûle hein. Et Monsieur le Ministre, je me tourne vers vous avec bienveillance mais exigence que tout dépend de vous. J'ai dit tout à l'heure en reprenant les propos de notre collègue Jérôme Durain qu'il y a la recherche de sens. Et la nécessité de sous entre guillemets parce qu'il y a une exigence de rémunération pour une fonction pivot, si on veut préserver la proximité communal donc Monsieur le Ministre, moi j'approuve votre idée de vraiment faire un travail de fond. Mais avec une échéance sur le nom il faut qu'il soit validé accepté mais faut que ça s'accompagne du 2ème volet c'est vraiment le sujet de la rémunération qui est d'un très grand sérieux. Monsieur le Ministre. Oui, je prends la parole maintenant parce que je pense qu'on est au fond au coeur du débat le sens la rémunération parcours recrutement les les les sujets ont été ont été bien posées. L'engagement il est pris. Et pas pour l'année prochaine pour travailler dans les prochaines semaines avec les employeurs territoriaux. Je l'ai dit à pouvoir aboutir sur ce chantier prendre date s'il doit y avoir un rendez législatif qu'on puisse le mener avant l'été et avoir un rendez-vous financier au moment du projet de loi de finances, comme cela a été proposé par le ministre Richard l'engagement. Est pris. Je je je tiens à dire ici aujourd'hui sur le nom vient d'avoir le débat. Les enjeux de rémunération. Bien sûr qu'il y ait un cadre de rémunération a fixé. Une réflexion indiciaire peut être qui doit être menée en parallèle de la fonctionner les actions du métier de secrétaire de mairie et des outils indemnitaire je veux juste dire essayer ne le prenait absolument pas comme quelque chose de quoi que ce soit de ma part mais il y a des possibilités indemnitaire qui existe aujourd'hui. Je les mentionne, vous le savez, il y a 4 Cadre d'emplois qui sont liées au métier de secrétaire de mairie juste mentionner le plafond du riz du Rifseep annuel brut qui est possible a engagé pour les communes aujourd'hui attachés territoriaux, 42.000 euros. Régime indemnitaire moyen, versé en 2019, 13.000 euros. Plafond Rifseep secrétaire de mairie en extinction. Vous l'avez rappelé 42.000 euros également. Régime indemnitaire moyen, versé en 2019, 3100 euros. Rédacteur territoriaux plafond du Rifseep annuel brut 19.860 euros. Régime indemnitaire moyen versant 2019 7700 euros. Adjoint administratif territoriaux plafond du Rifseep annuel 12.600 euros régime versé en 2019, 5400 euros. Donc je crois que ça mais aussi chacun face à ses responsabilités il y a un enjeu à fixer un cadre et que le gouvernement et c'est l'engagement que je prends aujourd'hui le fixera mais c'est la responsabilité partagée de l'ensemble des employeurs, dont les employeurs territoriaux et je dis ça sans rien minimiser les conséquences financières pour les employeurs territoriaux qui nous renvoie au débat budgétaire. Voilà, je voulais faire cette intervention peut être un peu synthétique. Pour la suite de nos débats. Pardon. Madame Varia cela. Enfin. Allons-y. je reprends l'amendement de de notre collègue Bourgi je que je partage totalement. J'ai fait ce métier toute ma vie, donc. Général puis ensuite. J'ai été DGS. Je pense que sur l'aspect formation. Déjà il faut savoir que. Pour avoir, pendant 15 ans. Formé des secrétaires de mairie, notamment sur l'élaboration du budget et la clôture des comptes. elles étaient particulièrement en difficulté à peine recruter il fallait faire le budget et vous savez c'est pas évident de faire un budget M. 14. Comme ça, de but en blanc et je pense que. Ce parcours de formation, il faut aussi prendre en considération que elle me le disait souvent quand elles viennent en formation elle fermer la porte de la mairie. Ça faut savoir que ça existe aussi et donc il faut. Organiser les choses de telle façon qu'elle puisse bénéficier de cette formation et puis je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Vous aviez laquelle la possibilité parce que j'ai suivi ce parcours vous aviez la possibilité il y a quelques décennies de préparer un diplôme qui était particulièrement intéressant. Certes, il fallait aller en cours du soir à la fac hein. Ce que je fis. Qui était le diplôme de l'École nationale d'administration municipale. Vous prépariez ce diplôme en en trois ans et puis ensuite vous prépariez le diplôme supérieur d'administration ne dit pas le des C'était des formations. J'ai beaucoup regretté qu'elle disparaisse parce qu'elles m'ont beaucoup apporté. Elle m'en a pris non seulement être. Tout à fait opérationnel dans mon métier. Elles m'ont permis de passer de gravir tous les échelons, puisque j'ai commencé par le concours de commis que j'ai continué par le concours de rédacteur et que je suis devenu à plus et DGS. Dans des villes beau très importante donc je regrette que ce parcours de formation n'existe plus et on ne devrait réfléchir peut-être

Donc évidemment les communes qui ont les moyens financiers. En plus la possibilité d'avoir des cadres de bon niveau, puisqu'elles offrent des intéressant que les petites communes. Décidément vous êtes plusieurs à profiter de ma bonté ce matin et je passe la parole au président d'Arnaud qui n'a pas connu les. Il était pas né. Mais monsieur le président d'Arnaud. Mais qui va continuer à abuser de votre bonté. Monsieur le Président, mais moins de deux minutes, je vous rassure. Simplement, je n'avais pas prévu d'ailleurs de de prendre la parole, mais suite aux propos du ministre on veut quand même réagir pour partager et adhérer aux propos que ma collègue vient de tenir et dire que Céline Brulin a raison. La sémantique, c'est important mais ce qui est important, c'est quand même la question de la rémunération et du salaire. Moi je viens d'un département aujourd'hui toutes les questions qu'on se pose on se se les pose même pas dans le même temps, on a plus de ressources humaines. Il y a quasiment plus personne parce que les communes sont très isolées très éloigné qu'il faut des moyens importants, notamment pour se déplacer, on on mutualise tant que faire se peut, mais ça reste quand même un sujet très compliqué le Rifseep tu sais très bien mais les communes dont je parle. Elles n'ont pas les capacités, j'allais dire d'abonder suffisamment et puis et puis parce que c'est le plus important c'est que ça reste des primes ça ne rentre pas dans le calcul pour la pour la retraite et qu'à un moment donné, au regard de l'expérience au regard de la valorisation. De ces femmes et ces hommes qui sont les chevilles ouvrières mais qui sont quasiment l'Alpha et l'oméga de la vie de nos communes. Je pense que c'est essentiel à prendre en compte et je pense Monsieur le Ministre, que c'est un chantier d'urgence. Je vous remercie. Oui, bien. Et voilà, Monsieur le Ministre, vous avez voulu lancer le débat. Le retour éclair plus de moyens pour nos communes. Alors après, vous vous débrouillez. Allez. Je vais mettre aux voix quand même l'amendement parce que l'air de rien on est là pour ça. Donc, l'amendement de 3 de Monsieur Bourgi avec 2 avis défavorables commission et gouvernement qui pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est rejeté, je mets aux voix l'article IV qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté à l'article 5. Une prise de parole monsieur Merci monsieur le président. Cet article vise à un soir la notion de promotion interne pour les secrétaires de mairie et c'est un élément particulièrement important est parti comment essentiel et je ne veux pas me faire l'écho de ce qu'on dit, nombre de nos collègues et fort justement par rapport à cela. Mais pour autant et je, j'vais déposé de deux amendements dans ce cadre-là il y a le 1er, essayer de faire mieux connaître. Cette profession de secrétaire de mairie et c'est là où le linge de stage et quelque chose d'essentiel pour des jeunes, pour qu'il. Il

un, un, un élément un élément essentiel. Mais il y a un autre point qui est une réalité et plusieurs l'ont dit et pour laquelle paraît essentiel que. Nous puissions la la la la prendre en compte. C'était le sens aussi d'un amendement que j'avais déposé. C'est. Cette notion relative au secrétaire de mairie qui exercent leurs fonctions dans plusieurs mairies dans des communes. Donc, et ce plus particulièrement. Pour celles pour lesquelles les mairies pour lesquels elle travaille sont à à des distances parfois éloignées et parfois elle travaille pour des demi-journées donc. C'est le matin dans une commune l'après-midi dans dans dans une autre et avec une allonge qui est parti quand même importante et je pense notamment et et peut être plus spécifiquement ou à celle qui travaillent en zone de montagne, pour lesquels c'est difficile et c'est compliqué et donc il nous apparaît essentiel aussi que dans le cadre des travaux de réflexion qui seront ceux du Sénat à la matière on puisse prendre en compte cet aspect. Des choses pour rendre attractive ses fonctions donc de secrétaire de mairie. Merci l'amendement quatre Monsieur Bourgi. C'est le même. Monsieur le. Président, Monsieur le Ministre, je vais faire mienne les sentiments de bienveillance et d'exigence de la présidente Françoise Gatel en vous disant, Monsieur le Ministre, j'ai pris acte de vos réponses. Je prends date du rendez-vous que nous aurons ici même et je retire cet amendement. Merci je mais aux voix l'article 5 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Je me vois l'article 5 bis qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté l'article 6 et supprimer l'article 7 est supprimé après l'article 7 l'amendement huit Merci monsieur le président. et pour moitié de représentants des agents administratifs représentant. Il émet des avis simple sur toutes les questions d'ordre général qui concerne ce Cadre d'emplois en fait par le biais de cet article c'est suite à des échanges que j'ai eu notamment et plus particulièrement avec Sylvian Calce qui le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale

les grandes communes et avec un cadre de fonction qui est totalement différent entre les grandes communes qui sont structurés avec des services et où le secrétaire général,

au regard de ce cadre et de ces éléments, par le biais donc de cet amendement. Il s'agit de mettre en avant ce cadre de spécificité et qu'il lui est ce cette instance j'allais dire d'échange et de dialogue à l'échelle départementale, qui pourrait être un élément important et et est essentiel. Comme je l'ai dit tout à l'heure et précédent manque. Le couple si vous voulez le duo secrétaire de mairie. Maire est un élément essentiel et là ce serait un cadre utile d'échange et de dialogue. Merci avait de la commission d'dans rapporteur. Merci Monsieur le Président et coûter cher collègue. Effectivement, vous vous pointez une une spécificité du métier de secrétaire de mairie. Cette fonction ne correspond plus un Cadre d'emplois unique à la différence des autres métiers de la fonction publique territoriale. Je suis d'accord pour dire qu'il y a un manque de visibilité. Mais pour autant. Votre amendement me semble poser plusieurs problèmes. Je vais essayer d'être assez explicite. Tout d'abord au centre de gestion, il existe déjà des représentants des agents de la fonction publique hein. Les représentants du personnel qui est qui émettent des avis sur les situations individuelles au collectif c'est seront les instances des C A P et le CST par exemple. Si une nouvelle instance paritaire été créé spécifiquement pour les secrétaires de mairie qu'elle serait sa place et quel serait son rôle par rapport justement aux instances que je viens de citer. Ensuite les cendres de gestion n'ont pas de compétence particulière pour gérer une instance qui émettrait des avis qui concerne l'ensemble d'une profession, il me semble. Il a d'autres institutions comme le, le, c'est le, le Conseil supérieur de la fonction publique qui pourrait être plus à même. D'abriter en leur sein une une instance. Du type que que celle que vous prévoyez ensuite l'amendement est insuffisamment précis. La mesure ne serait donc pas opérationnel ne sont prévues, ni les modalités de désignation des membres ni les modalités de fonctionnement de l'instance ni le sort réservé aux avis qu'elle pourrait émettre. Et enfin. De façon plus singulière, l'instance. Que vise à créer votre amendement émettraient des avis pour plusieurs Cadre d'emplois mais uniquement pour des fonctions particulières ça poserait un problème d'égalité vis-à-vis des autres Cadre d'emplois. Des des autres cadres, membres de ces mêmes cadres d'emploi. Donc vous voyez pour toutes ces raisons je vous demanderai le retrait sinon un avis défavorable.

Merci monsieur le président. issus des collectivités locales et des représentants donc des secrétaires de mairie. En fait, cela a été dit par nombre de nos collègues au regard donc de la. De la classification par âge des secrétaires de mairie nombres d'entre elles vont partir à la retraite dans les années à venir et que donc il y a lieu d'anticiper par rapport à cela et en liaison donc avec. Les représentants dans des collectivités, il s'agit d'essayer de mettre un cadre pour essayer de

entre élus et et entre représentants des des des secrétaires de mairie et notamment je le dis par rapport à cette association nationale qui est en train de se structurer, de secrétaire de mairie. Il y a déjà un certain nombre de départements. Donc où où elles sont implantées. Il y en a d'autres sur lesquels c'est en train de se faire et je crois que c'est. Un point important d'autant plus qu'elles sont particulièrement et pour répondre à votre interrogation. Madame la rapporteure tout à l'heure les CRP sont dans un cadre et qui sont plutôt pour traiter des schémas individuelle dans la réalité du terrain. C'est ce qui se passe et ce que je propose au travers de ces amendements qu'il y ait un cadre un petit peu plus collectif pour des enjeux qui sont des enjeux spécifiques par rapport à ceux des secrétaires de mairie et qui ne seront bien sûr pas forcément soluble dans les dans les autres éléments puisque c'est ce que nous l'avons dit et les uns et les autres depuis, depuis ce matin les secrétaires de mairie. on et exerce une fonction particulièrement singulière et qui mérite d'être traités comme telle. Merci Monsieur le Président, simplement monsieur Folliot pour répondre à votre dernière interrogation. Vous avez raison, laisser happer traite des des des sujets individuel mais le CST traite des sujets collectifs et à l'intérieur d'insister peut tout à fait y avoir. Un groupe de travail

ainsi et je pense aussi au Conseil supérieur de la fonction publique. Mais pour revenir à votre amendement. Vous avez là aussi encore raison il y a effectivement de, de grosses difficultés pour le recrutement. Alors je vais encore par les descentes de gestion. Ah parce que vous savez quand même que c'est le tiers de confiance privilégié des communes et notamment des communes rurales qui doivent s'appuyer vraiment sur sur leur service, et actuellement les centres de gestion ont la possibilité de mettre à disposition. Des agents pour remplacer les secrétaires mairie quand elles, elles vont en formation et je pense qu'il y aura un partenariat encore en plus à développer, ils le, ils Ils n'ont pas forcément toujours bien les moyens mais je sais qu'il y a beaucoup de sortes de gestion qui sont en train de recruter spécifiquement des agents au niveau secrétaire de mairie ou de les former pour ça justement pour répondre aux attentes particulières des des collectivités. Ne pas oublier que les petites collectivités. Il y a pas de c'est pas péjoratif de ma part sont vraiment le coeur de métier et d'attention des des de gestion. Donc je crois qu'il faut vraiment leur faire confiance pour donc soit. des des des remplacements soit embauché des itinérante et les mettre aussi à disposition donc très sincèrement un conseil adopte pour pour. Trouver une solution. Ça me paraît pas très très adaptée très adéquat. Donc je vous demanderai là aussi le retrait ou un avis défavorable je suis désolé. Avis du gouvernement, en tous points le même avis que Madame la rapporteure de ces primaires ses. Demandes de parole, monsieur Villach. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Moi aussi j'ai suivi la formation du des C'était il y a très longtemps, je ne vous le cache pas. Et puis j'ai. Également. En qualité de président de centre de gestion. Déléguée. FPT met en place des formations initiales de secrétaire de mairie.

parce que c'est ça qu'il faut qu'on, c'est la solitude du secrétaire de mairie. Et oui les seuls, hé bien c'est un vrai défi à surmonter parce que il y a tant de sujets traiter Tan de compétence à maîtriser tant de dossiers à connaître que c'est quasiment impossible même avec le fromage. je n'ai pas déposé l'amendement parce que je pense que je suis à l'autonomie, je ça relève plus du réglementaire. En. 98 ma secrétaire de mairie lorsque j'étais maire ma. Informé de son le fouet là partir à la retraite à de 2000. Et à ce moment-là, il existe des dispositifs qui s'appelait les emplois jeunes. Et donc j'ai recruté une personne en emploi jeune largement prises en charge par l'État. Et cette personne pendant 3 ans elle a continué sa formation, elle avait déjà un DEA d'administration mais la perfectionner sa formation pratique sur les communes et a même autant auprès de l'ancienne se mérite secrétaire le mairie qui partent à la retraite. Elle a pris le côté pratique à la maîtriser. Toutes les difficultés quotidiennes et je dois vous dire qu'en 2001 comme secrétaire de mairie à partir alors je travaillerai avec elle depuis 20 ans. Ça m'a fait un peu de peine qu'elle parte mais au niveau du fonctionnement de la mairie et le fait rien passé parce que j'avais quelqu'un qui est depuis 3 ans en prenez le métier sur le tas énorme je le ministre, je vous propose de réfléchir à ça. Des recrutements de contrats aidés. Monsieur le président, Monsieur le Ministre. Quelques éléments de réponse à notre collègue Folio sur cette instance de répartition. Je n'en suis pas convaincu, vous le savez se pose souvent la question pour l'installation des médecins libéraux pour lutter contre la désertification médicale et les mêmes arguments que nous entendons ici sur l'absence de coercition possible. Je ne vois pas de quelle façon. De quelle manière, avec quels outils on pourrait répartir de manière autoritaire au coercitives secrétaire de mairie. En revanche, une information que je voulais verser à votre connaissance dans le cadre de la région Occitanie. Nous avons mis en place une expérimentation avec l'Association des maires de France qui a la mission de recenser auprès de tous les maires du département, la secrétaire de mairie qui partent à la retraite ou qui vont connaître des changements de postes pour des raisons de mutation, ce qui fait que lorsque nous mettent en place les formations initiales. Pour les personnes qui sont sélectionnés par Pôle emploi à la fin de la formation, nous leur remettons une liste de communes de plusieurs dizaines de communes qui ont besoin à l'instant-et d'un secrétaire de mairie parce qu'il y a un poste vacant aux des mairies qui dans les semaines ou les mois qui viennent, auront besoin d'un secrétaire de mairie, ce qui permet aux candidats d'identifier territoire par bassin territorial à l'intérieur du département mais parfois aussi sur des départements voisins et sur les territoires mitoyens vers lesquels. Et en tout cas, ça permet d'atteindre la répartition équitable sur le territoire et surtout la plus efficace et la plus efficiente possible parce qu'il y a le frein de la mobilité. Un secrétaire de mairie qui habite dans le département de l'Hérault mais qui, à la frontière avec le département de l'Aude en frontière à la frontière avec le département du Tarn qui vous est très cher cher collègue pourrait postuler sur votre département et il n'y a pas de cloisonnement administrative entre nous. Je mais aux voix l'amendement 10 avec 2 avis négatifs qui est pour.

Oui, monsieur le président pour une explication de vote sur sur ce texte pour déjà remercié le groupe CRCE d'avoir proposé cette ce texte pour remercier la Commission du, du travail. Fait. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de rendre hommage à l'action de ses secrétaires de mairie qui sont des véritables piliers de notre action communale de Rita, petites mains de de la République. Et. Je veux dire. y a beaucoup d'initiatives locales très intéressante, qu'il convient. De pouvoir démultiplier. Ça a été signalé par par le rapporteur. J'ai en tête, notamment dans l'Yonne. Ce qui se fait avec l'Asie Hamas qui est l'association de secrétaires et employés administratifs des maires de l'arrondissement de sens qui permet de de croiser les regards de d'échanger les expériences et indéniablement, il y a un besoin d'extension de ce type de dispositif parce que il y a pas un maillage intégral du département, je dois le dire et je pense que c'est pas un cas unique. En France, et puis c'est important à travers ce texte de de conforter l'évocation l'attractivité de cette mission de ce métier parce que ayant aussi en tête que les secrétaires de mairie d'aujourd'hui hé bien ce sont souvent les élus de demain. Il se trouve que j'ai fait mes gammes de conseiller municipal à Valérie sous l'égide de Dany Cerdain mère qui fut longtemps, 16 ans, secrétaire de mairie de la commune. J'ai aussi en tête Isabelle Poulin, maire d'éclairer moi qui pendant 41 ans, a été secrétaire de mairie à Fontaine La Gaillarde, si vous dire que nous avons là aussi un vivier de femmes et d'hommes qui. Sont tous prêts à s'engager et et je me réjouis que avec ce texte, ça a été dit, c'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Il y a des dispositions pour la formation, il y a des dispositions pour l'avancement. Le travail va se poursuivre. Il y a les sujets indemnitaire il y a des sujets de dénomination. Et je me réjouis que nous puissions continuer avec la mission d'information avec peut-être des éléments en loi de finances et surtout l'engagement plein entier du ministre dont je sais l'attachement à réussir ce chantier et le mener à bien, je vous remercie. Merci madame Darcos. Oui merci président. Moi aussi je voudrais à mon tour saluer l'initiative de notre collègue Céline Brulin, et et notre rapporteur, je suis très heureuse qu'on puisse en en effet voter tout ce texte. On rend hommage aujourd'hui à des, des femmes et des hommes qui font vraiment le, le ferment de nos, de nos petites communes et ça a été dit par plusieurs personnes. Monsieur le Ministre, elles ont souvent la tâche difficile. Au-delà d'avoir des relations humaines très important et de former un tandem très fort avec leur mère. De devoir remplir des dossiers extrêmement complexe de demande de subventions en ce moment on est dans les commissions DETR. Autres. le gouvernement nous a beaucoup vendu le fond Vert c'est encore des études encore des des manipulations très complexe. Une de mes collègues parler de remplir des dossiers fédère il y en a pas beaucoup qui arrive à le faire mais même des contrats territoire et ce sont donc des gens à qui on met une pression énorme pour aider les mères à remplir ce genre de, de dossiers et je sais que lorsqu'il y en a un qui y en a qui manque. Il y a une solidarité, mais évidemment qui se crée. Moi j'ai été le l'autre jour dans une mairie où justement leur manque une depuis quasiment trois, quatre mois. Les autres communes d'à côté se solidarisent pour essayer de lui prêter main forte. Mais, mais c'est vrai que c'est vraiment. Un poste tellement crucial qu'il faut les aider. Donc aujourd'hui on leur rend hommage à travers votre loi chers collègues et et j'en suis vraiment heureuse. monsieur le président. Monsieur le Ministre, madame la rapporteure. Je tiens également à féliciter les sénateurs du groupe communiste d'avoir attiré l'attention à juste hauteur sur ce métier magnifique et indispensable et très rapidement je tiens à apporter aussi un témoignage de l'expérience de l'expérience de la communauté de commune Mademoiselle dans ce domaine avec 50, petite commune un service mutualisées de secrétariat, a été mis en place il y a 10 ans, il concerne aujourd'hui. 30 communes qui n'ont plus de problèmes d'attractivité. Dans ce métier, bien au contraire. C'est à l'initiative de son DGS très créatif, le Vosgien Jean-Charles De Belie qui a été mis en place ce dispositif, de même qu'il a été créé avec le Centre de gestion hein DU qui a un taux d'insertion professionnelle qui dépasse les 90%. Ils ont maintenant une idée assez originale que je tiens à vous présenter celle d'une mairie virtuel à l'échelle de ces 50 communes en plus du présentiel. Il s'agirait par un numéro unique et un site internet unique de pouvoir répondre aux concitoyens du lundi au samedi, de 8h du matin à 8h du soir et je pense que c'est une initiative extrêmement intéressante qui mériterait, Monsieur le Ministre, d'être encouragé, je vous remercie. vous remercier par avance du vote qui semble se dessiner dans cette assemblée, remercier la rapporteure avec qui je crois, nous avons travaillé en confiance et en loyauté. Dire et je crois que nous sommes tous en phase là-dessus aussi que l'adoption de cette proposition de loi est en effet un point de départ d'un travail et vous le dites vous-, même monsieur le maire qui doit se poursuivre sur. Des champs, on le voit assez vaste, on a évoqué la formation je n'y reviens pas, si ce n'est pour pointer ce qu'on dit fort justement les collègues. C'est-à-dire que. La formation, les secrétaires de mairie aujourd'hui la font sur leur temps libre ou en fermant la porte de la mairie et que ça c'est un sujet aussi à part entière qu'il faudra traiter revenir peut-être pour qu'on ne se méprenne pas, Monsieur le Ministre, sur, effectivement, c'est un véritable métier. Mais le statut de la fonction publique est aussi très fécond et ça n'est pas nous qui sommes les modestes continuateur. De d'Anicet Le Pors, un de vos illustres prédécesseurs, qui allons dire ici le contraire. Françoise Gatel a a dit. Qu'il fallait attirer et fidéliser une autre collègue a dit les élus passent mais les secrétaires de mairie reste. Et donc on voit bien que le statut. Dans ce qu'il a de meilleur peut permettre cette fidélisation et même ces évolutions de carrière et enfin. Je voudrais revenir et prendre date clairement avec vous, vous avez évoqué après qu'on faisait interpeller le prochain PLF. Je crois que me faire la voix de tous ici pour dire que nous prenons date pour que des mesures significatives puissent être prises au prochain PLF il faut regarder avec Intelligence. Comment. Mais d'ores et déjà. La piste de la bonification indiciaire doit être explorée. On l'a évoqué 15 points de plus depuis un an, 15 points de plus et 70 euros c'est même pas si je peux le dire de manière triviale, un plein d'essence aujourd'hui quand on sait que les secrétaires de mairie doit faire des kilomètres par semaine pour se rendre d'une mairie à l'autre, elles exercent donc voilà des pistes qu'on continuera à travailler ensemble et je pense que c'est cette adoption va être un 1er plan d'appui. Merci Oui, merci monsieur le président. Je suis président de la Commission, monsieur le ministre, madame la rapporteure. Juste quelques mots effectivement pour se, se féliciter de de la situation, puisque grâce. À cette proposition de loi. Le sujet sur la table et on a vu qu'il avait déjà un certain nombre de de consensus un consensus pour rappeler que la fonction, le métier de secrétaire de mairie était un était une fonction essentielle à notre territoire et qu'il appartenait aussi à l'État en lien avec les collectivités de s'assurer de l'administration dans l'ensemble de de nos collectivités dans l'ensemble du territoire et donc de de permettent de faire avancer ces sujets de. Deuxièmement qu'il y avait un consensus sur le fait que. Il fallait prendre à bras le corps ce problème et qui avait des, des solutions. Qui, qui devait être trouvé certaines et la plupart seront probablement d'ordre réglementaire, un consensus sur le fait que c'est un vrai métier. C'est pas une fonction qu'on comme comme une autre, c'est un vrai métier, c'est un beau métier qui a tous les atouts pour être attractif, puisqu'il est polyvalent. C'est un métier de contact, c'est un métier de où on trouve des solutions. C'est un métier qui n'est pas uniquement admnistrative qui est aussi un métier stratégique à l'instar du maire, c'est le seul métier où on participe. Aussi activement à la vie de de la commune et notre territoire et donc pour cela. Il faut qu'on puisse avancer, qu'on puisse travailler à la fois sur la reconnaissance de ce métier dans ces différentes formes le statut. La formation évidemment une formation peut-être moins académique que celle qu'on arrive à proposer aujourd'hui une formation qui soit pratique sur les gestes du quotidien, c'est ça qu'attendent vraiment les secrétaires de mairie une formation beaucoup plus pratique, un accompagnement puisque c'est quand on est confronté au problème qu'on a besoin. Des fois d'avoir une solution et pas forcément dans une formation initiale académiques et dans les conditions de travail d'ses secrétaire de mairie. Les sujets sont sur la table aujourd'hui, il va falloir qu'on, qu'on s'y penche. Avant de refermer le dossier. C'est un enjeu majeur pour la vie de nos territoires ruraux. Et Madame Cukierman. presque intrinsèques au fonctionnement de la vie communale qui représente ses secrétaire de mairie sur le président, vous l'avez dit, avec une petite pointe d'ironie tout à l'heure dans dans dans vos propos mais je crois qu'au-delà de l'ironie, c'est une réalité. Monsieur le Ministre, bien évidemment, nous le disons il y a besoin de continuer de travailler, il aura besoin des financements à la hauteur. Nous ne voudrions pas ici et je crois collecte le dire de façon très collective, donner le sentiment que, en améliorant la qualité et le statut et les revenus des secrétaires de mairie cela aurait demain des confidents Graves pour les finances communales et c'est donc bien un ensemble. Donc vous nous l'avez dit et vous nous y avait invités. Nous nous retrouverons. Au prochain projet de loi de finances certainement avance je je n'en doute pas sur d'autres sujets, mais en tout cas sur ce point très précis d'ici là, la délégation aux collectivités territoriales. Cela a été évoqué et plus particulièrement notre collègue Cédric Vial sur ce point précis des secrétaires de mairie aura je n'en doute pas avancer. Et donc nous avons d'autres rendez-vous pour continuer de faire avancer cette réflexion, c'est un, un point de départ je crois qu'en tout cas c'est une volonté que nous avions avec ma collègue Céline Brulin, au moment de l'élaboration de cette proposition de loi. Tout d'abord, pas simplement une reconnaissance mais une prise en compte faire entrer dans toutes nos réflexions que ces personnes souvent de longs parfois que l'on ne. Qu'on ne met pas suffisamment en avance, si ce n'est pas la distribution de médailles. En tout cas sont fondamentales et que cela méritait bien un temps de travail législatif et je veux vraiment remercier Madame la rapporteure pour avoir permis permis aussi que nous puissions en arriver jusqu'ici ce matin elle comprendra bien évidemment à travers les collaborateurs de la commission des lois. Ce que je veux dire par là. Merci pour. Merci. Je vais mettre aux voix donc la proposition de loi visant à revaloriser le statut de secrétaire de mairie qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Elle est adoptée à l'unanimité. Écoutez je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre. Je vais m'adresser maintenant au groupe CRCE. Vous êtes dans votre niche et il y a le 2ème texte on le démarre, c'est une heure et demie. Le texte, mais si on le démarre. Ça veut dire que on essaye de faire parce que on ne peut pas le découper en morceaux, on essaie de faire jusqu'à l'intervention d'Alain Ministre, c'est-à-dire en gros jusqu'à 1h13 On est d'accord. Ah vous reprendrez après mais par définition. À 14h 55. Voilà on est d'accord. Hé bien alors c'est parti. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative à la maîtrise de l'organisation algorithmique du travail présenté par Monsieur Pascal Savoldelli Madame mesdames Katia pour se Laurence Cohen et plusieurs de leurs collègues. Dans la discussion générale. La parole est à monsieur Pascal Savoldelli, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes.

Monsieur le Président Madame la Ministre. Mes chers collègues. Avant de commencer. Je tiens à saluer les mobilisations sociales qui se tiennent partout en France aujourd'hui. Parce qu'en réalité les enjeux de cette réforme des retraites et sur l'uberisation sont très liés. D'ailleurs je vous le rappelle, mes chers collègues, que si les travailleurs des plateformes été requalifiée en salariés ben il permettrait de rapporter 1,45 milliards d'euros à la Sécu et son régime de retraite par leurs cotisations. Cette proposition de loi que nous présentons aujourd'hui avec notre groupe communiste républicain citoyen et écologiste s'inscrit, vous le savez dans le prolongement de plusieurs années d'engagement aux côtés d'acteurs sociaux, syndicaux universitaires et politiques mobilisés aux côtés des travailleurs et travailleuses des plateformes numériques de travail avec mon collègue Fabien Gay. Nous avions déjà au sein du collectif Pédale et tais-toi, rencontrer des livreurs en France qui nous avez décrit la réalité mais j'irai dire surtout la précarité de leur situation. Il faut qu'on s'entende, là on parle de travailleur dit. Indépendant. Mais qui sont dépendants économiquement. Cette précarité est le fruit d'un modèle économique celui du capitalisme de plateformes dont le coeur de l'action repose sur un contournement des règles notamment du droit du travail mais aussi de la concurrence par le biais du management algorithmique. Ce modèle économique qui entraîne un retour au temps d'avant. Le contrat de travail. Ou les risques reposait uniquement sur les travailleurs lorsqu'il n'avait aucun pouvoir et où les normes sociales n'existait pas en misant sur le concept d'indépendants ah fausses statues. Les plateformes numériques recrée l'organisation et la rétribution du travail à la tâche, grâce à un management algorithmique que je qualifie de brutale et d'injustifiable. Mes chers collègues. À l'heure où nous ne pensons plus le travail qu'au prisme de la valeur qu'il produit. Il est temps de faire le point sur les coups de cette production. Ces coups, il s'appelle Franck page 18 18 ans étudiant et coursier pour UberEats ce soir-là il livrer un repas à vélo lorsqu'il fut renversé par un camion avant de trouver la mort. UberEats estime que ce décès n'est pas de sa responsabilité. Un dramatique accident de la route mais pas un accident du travail. Pourtant cet itinéraire lui avait été imposée par la boîte noire l'algorithme ce même algorithmes qui le menaçait de le déconnecter s'il n'allait pas assez vite. Il s'agit ici d'un exemple de coursiers une figure parmi les plus visibles de l'uberisation. Pourtant ce modèle touche à tous les ports de l'économie, le transport, les services à domicile ou encore les micros travailleurs du clic ces tâcherons qui se trouve parfois à l'autre bout du monde aussi pour réaliser des micro-tâches invisibles pour dire entraîné la machine. Mes chers collègues ce management désincarné. Déshumanisé doit cesser. Il s'assoit sur la loi et sur le droit des travailleurs le flou de l'algorithme qui attribue les commandes évalue leur réactivité, calcule le parcours et le temps de trajet réalisé ce même flou qui agit comme une épée de Damoclès au sud la tête des livreurs, les poussant à aller toujours plus vite qui en laisse le choix aux livreurs que la pression de la déconnexion brutal et injustifiable ce flou rythmé par l'injustifiable. Un flou rythmée par l'immédiateté allez peu importe la sécurité et le bien-être de celui ou celle que l'on note d'une ou plusieurs étoiles au gré de nos services. La boîte noire de l'algorithme n'est pas un simple outil dénué d'intentions politiques. Elle est le fruit de décisions de ses fondateurs qui oriente les comportements des travailleurs inscrits sur ces plateformes. Le management algorithmique constitue de fait pour de nombreuses plateformes numériques de travail, un outil de contrôle de direction de sanctions le travail que nous avons porté collectivement au sein de la mission d'information. Va également dans ce sens dans le rapport qui en est issu. Fruit d'un travail de plus de 3 mois avec notre collègue la sénatrice Martine Berthet et grâce à l'audition de plus de 60 acteur ce rapport voté à l'unanimité a permis la la formulation de plusieurs recommandations portant sur la nécessité de mieux réguler mais aussi d'exiger davantage de transparence des algorithmes de ces plateformes numériques de travail. Je prends pour exemple la recommandation numéro 9. Qui fait partie des recommandations qui ont été votées à l'unanimité. Je la cite, engager une réflexion pour adapter le droit du travail aux spécificités du management algorithmique et à ses conséquences sur les conditions de travail. Alors que l'algorithme est devenu le contremaître des temps modernes. Il s'agit de rattacher la décision algorithmique à Lourdes patronale et, contrairement aux discours des plateformes l'algorithme n'est pas un outil neutre. Qui serait dépourvu de subjectivité. Une décision qu'on prend toujours une part de subjectivité, même lorsqu'elle est autobaptisés il subsiste donc un risque de standardisation de critères de gestion du personnel mais également un risque de discrimination. Si on intègre dans un algorithme le sexe, l'âge ou encore le lieu de résidence ou je ne sais quel autre critère. Cette présente, proposition de loi propose donc un nouvel angle d'attaque. À la requalification du statut des travailleurs des plateformes numériques. En effet il faut savoir qu'aucun texte aujourd'hui aucun texte de droit public, ni de droit privé. Ne défini à proprement parler la notion de salariat. Ce statut découle directement de la relation de subordination qui en est constitutive, c'est pourquoi cette proposition de loi tend à mettre à jour la relation de subordination existante entre l'algorithme. On pourra appellent de leurs d'ordres et le travailleur ou la travailleuse de la plateforme numérique. Il est extrêmement important devrait vers l'ouverture de la boîte noire de l'algorithme son opacité et problématique et en particulier pour les travailleurs et travailleuses concernées rapport du défenseur des droits et de la et de la CNIL datant de mai 2020 alertait déjà sur cet angle mort du débat public. Les exemples de dérive et de discrimination par le biais des algorithmes sont nombreux et sur une grande diversité de plateformes différentes, on a eu des cas par exemple de déconnexions abusives chez les plateformes comme Deliveroo suite à des mobilisations sociales pouvant ça pas rater s'apparenter à la répression syndicale, comme cela avait été documenté par Cash Investigation ou encore de discriminations femmes-hommes à l'embauche chez Amazon. Et ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres, l'un des leaders de la lutte des chauffeurs VTC Brahim Ben Ali nous disait hier que le discours du beurre pour répondre à leur demande d'une plus grande transparence algorithmique consistait à leur répondre, je les cite, on ne va pas vous donner le secret de notre algorithme. Ce serait comme donner la recette de Coca Cola. D'accord mais le secret des affaires peut pas contourner hein nécessaire encadrement quand il touche aux conditions de travail et au risque de discrimination. Nous ne parlons pas là d'une boisson. Nous parlons de vies humaines de centaines de milliers de travailleurs et travailleuses. Nous allons vers la fin de la hiérarchie du salariat, tout en maintenant une subordination accrue et renouvelées dans l'esprit de la start-up chacun devient son propre employeur une entreprise d'ailleurs de soi. Eh bien posez-vous la question, où est l'utilité sociale d'un travail. De quoi parle-t-on avec la valeur travail et je dirais même de la valeur humaine. Alors, mes chers collègues, ne faisons pas comme les avions, n'attendons pas que l'avion se crashe pour ouvrir la boîte noire l'algorithme type Uzi moins qu'un contrat de travail mais un contrat, dont les premiers concernés n'ont pas accès aux informations les plus fondamentales qui concernent directement leurs conditions de travail. Les travailleuses et les travailleurs des plateformes numériques ont pourtant besoin de code source, autrement dit d'être informé de l'intervention humaine qui se trouve à la source de la subordination à cet ordre algorithmique cette machine qui décide à quel moment vous êtes rentable en faisant de ces travailleuses et ces travailleurs des tâcherons corvéables à merci. L'algorithme c'est aujourd'hui investi dans tous les pans de notre société, qu'il s'agisse de Parcoursup pour les étudiants, avec tous les problèmes de sélection qu'il a pu poser ou encore la sélection de dans les cadres dans le cadre de recrutement dans certaines entreprises, dont la sélection fait parfois preuve de discrimination. Il est donc crucial. De regarder de près ce qui s'y passe, c'est tout le sens de cette proposition de loi ainsi l'article indéfini la Gorrite sur le plan juridique comme pouvoir de direction et de contrôle lorsqu'il joue un rôle de subordination d'un employeur ayant un impact sur ses employés. L'article de notre proposition de loi engage la responsabilité de l'employeur en prévoyant l'obligation, pour ce dernier de démontrer que l'algorithme n'est pas source de discrimination et l'article 3 précise la différence entre une simple plateforme de mise en relation et une plateforme jouant un rôle effectif d'employeur. Notre projet de loi propose humblement. De maintenir ouvert le débat sur cette question sans prétendre pour autant être la réponse à tout. Il s'agit avant tout de maintenir le débat ouvert sur le plan national, car nous savons que le projet de directive européenne sur cette question va dans le même sens, cette directive constitue une belle avancée pour les droits des travailleurs des plateformes confirmant une présomption de salariat et permettant de lutter contre le travail dissimulé et nous nous la défendons pour autant la France se pose davantage comme un défenseur aujourd'hui encore des lobbies des plateformes. On a témoigné l'affaire en témoigne encore l'affaire Hubert Fayard. Nous devons maintenir la pression car ce management algorithmique. Est aujourd'hui le plus grand cheval de Troie néolibéral qui finira par s'inviter dans toutes les formes de management au travail donc je vous invite fortement mes chers collègues à voter cette proposition de loi. fois premiers cette proposition de loi la frappe. À reconnaître les droits des travailleurs des plateformes avant même la fin du processus législatif européen. Cette proposition de loi constitue un nouveau jalon important vers un chemin qui reste encore long pour protéger à la fois les travailleurs et les travailleuses des plateformes mais également et je tiens à le dire également pour protéger les entreprises et les commerces qui sont en proie à une concurrence déloyale du point de la part des plateformes numériques de travail, tout cela, il faut respecter les règles du jeu donc oser Ozon lui donner les moyens d'accomplir son objectif. Donc évidemment, je vais vous dire que je vous appelle à fauté. Cette proposition de loi. Merci de votre attention et surtout à ceux qui sont présents. Merci. Collègue, la parole est maintenant Madame Katia pour se rapporteur de la commission des affaires sociales pour 10 minutes. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues, la surveillance constante l'évaluation permanente des performances l'application automatique des décisions sans intervention humaine. L'interaction des travailleurs avec un système et la faible transparence des algorithmes, tels sont les éléments constitutifs du management algorithmes selon le Bureau international du travail. La proposition de loi de notre collègue Pascal Savoldelli qui travaille avec Fabien Gay depuis plusieurs. Années des membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. À bord de cette réalité. L'utilisation de l'algorithme pour l'organisation du travail et la gestion de la main-d'oeuvre déjà bien présentes dans le monde du travail. Elle est pourtant ignorée de notre droit. L'apparition des plateformes numériques a entraîné une rupture technologique en permettant à une multitude d'acteurs, d'être mis en relation en temps réel. Elle a aussi initié un bouleversement de l'organisation du travail par le recours à des algorithmes dans les secteurs des VTC de la livraison de marchandises en véhicules à 2 roues. Les travailleurs quoique formellement indépendants sont soumis à un degré élevé de contrôle et à une nouvelle forme de dépendance. Même s'ils peuvent choisir de se connecter ou non à l'application et à quel moment ils le font, ils sont en réalité privées d'autonomie dans la réalisation de leurs prestations. Ces travailleurs précaires et contraint de recourir à des formes à ces formes d'emploi cumulent les fragilités faibles revenus protection sociale incomplètes, absence de garanties en matière de temps de travail et de droit au repos forte Exposition aux risques professionnels isolés, ils sont de surcroît ni en compétition permanent par les algorithmes. Ces derniers apparaissent dès lors comme des boîtes noires sur lesquelles les travailleurs n'ont aucune prise ni aucune visibilité. Cette. Plateforme nisation. De l'économie se généralise à l'ensemble du monde du travail les algorithmes sont déjà de plus en plus utilisée pour gérer les ressources humaines au sein des entreprises. Intervention dans le processus de recrutement, la gestion des évolutions de carrière ou l'évaluation des salariés des logiciels peuvent ainsi analyser et comparer les comportements des candidats lors d'entretiens de recrutement si elle permet des gains de productivité cette gestion algorithmique du travail est porteuse de risques de surveillance abusive et généralisé de perte d'autonomie et de discrimination accru le sentiment d'aliénation qui peut alors gagner les travailleurs et facteurs de risques psycho-sociaux en outre cette gestion algorithmique tend à déresponsabiliser les employeurs et à priver les acteurs du dialogue social de leur rôle en matière de détermination des conditions de travail. Les risques sont d'autant plus important que le fonctionnement des algorithmes peut échapper aux employeurs eux-mêmes qui ont souvent recours à des solutions technologiques développées en externe dans son rapport du 29 septembre 2001 sur l'uberisation de la société. Pascal Savoldelli, à considérer qu'un algorithme n'était pas seulement une suite d'opération permettant de traiter des volumes importants de données mais bien une chaîne de responsabilités humaines. Quel que soit son degré d'automatisation la gestion algorithmique engage la responsabilité de personnes auxquelles il devrait être possible de se référer. Il a ainsi préconisé d'adapter le droit du travail aux spécificités du management algorithmique et à ses conséquences sur les conditions de travail. La proposition de loi traduit cette conviction afin de reprendre le contrôle de l'organisation algorithmique. Certes les algorithmes constitue une aide considérable pour améliorer l'organisation des entreprises et exonérations les exonérer les travailleurs de tâches parfois répétitives et contraignant. Toutefois, lorsqu'ils sont utilisés à des fins d'organisation du travail. Il devrait toutefois être encadrée et contrôlée, ainsi les travailleurs devraient être informé de l'utilisation de ces outils et avoir accès à leurs modalités de fonctionnement dès lors qu'ils affectent leurs conditions de travail. Quant à l'employeur il doit demeurer entièrement responsable des décisions qu'il prend dans l'entreprise. L'utilisation d'algorithmes devrait être considéré comme un simple outil d'aide à la décision. L'article premier inscrit donc dans. Donc les décisions des employeurs prises à l'aide de moyens technologiques. Parmi les décisions relevant de leur pouvoir de direction ils renforcent l'accessibilité du contenu des décisions. L'information du salarié sur les motivations des décisions le concernant et lui permet de demander qu'une nouvelle décision soit prise par un être humain. Par ailleurs, l'article de vise à assurer le respect du principe de non-discrimination dans l'utilisation des algorithmes. Par les tripes qu'ils opèrent et les recommandations qu'il formule en fonction d'un ensemble de critères les algorithmes peuvent conduire à des discriminations, des travailleurs contraires à la loi. Celle-ci peuvent même survenir indépendamment de la volonté de l'employeur. Une telle situation s'est déjà produite en 2017 l'entreprise Amazon a dû renoncer à l'utilisation d'un algorithme pour le recrutement de salariés car il induisait une discrimination à l'embauche en privilégiant les hommes aux femmes. Le logiciel s'appuyer sur une base de données recensant les CV reçus par l'entreprise depuis 10 ans, qui comprenait une grande majorité de CV d'hommes l'algorithme en a déduit que les candidats masculins était préférable et rejeté les candidatures féminines. Face à de tels risques. L'employeur doit être responsable des outils technologiques qui l'utilise pour le recrutement ou la gestion des salariés dans l'entreprise. La protection des travailleurs contre toutes les formes de discrimination au travail ne saurait être affaibli par l'utilisation d'outils technologiques pour l'organisation C'est pourquoi l'article de pose le principe selon lequel en cas de litige, l'employeur doit apporter la preuve que les outils qu'ils zut qui l'utilisent, ne sont pas source de discrimination. La proposition de loi s'attache enfin à mettre en lumière la situation des travailleurs plateforme qui est le résultat le plus visible de l'influence des algorithmes sur le monde du travail. excusez-moi juridique de ces travailleurs dont le Sénat a déjà eu l'occasion de débattre à plusieurs reprises est une question d'ordre public social. L'ambiguïté de leur situation lorsque l'algorithme de la plateforme joue un rôle essentiel dans l'organisation du travail donne lieu à un contentieux abondant auquel la réponse des juridictions n'est pas univoque. Plusieurs décisions de la Cour de cassation pencher dans le sens de la requalification salariés de livreurs à vélo de chauffeurs de VTC mais elle non. Pas une portée absolue. de la prestation de service et fixe son prix. Elle a une responsabilité sociale à l'égard des travailleurs indépendants, recourant à ses services, en particulier la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et les ordonnances du 21 avril 2021 et du 6 avril 2022 ont posé le cadre d'un dialogue social entre travailleurs indépendants et plateformes dans le secteur de la mobilité. Les premières avancées obtenues dans ce cadre ne sont pas négligeables. Toutefois les droits. Spécifiques progressivement accordée à ces travailleurs ont surtout eu pour effet de les enfermer dans un statut d'indépendant améliorer et de conforter le modèle des plateformes qui repose sur le contournement du droit du travail et le dumping social. Ses réponses à l'uberisation ne sont donc pas à la hauteur le statut d'indépendant n'est pas adapté à la situation des travailleurs précaires, qu'ils soient livreur à vélo ou chauffeurs de VTC et ne correspond pas à la réalité des relations entre ces travailleurs et les plateformes si le même débat existe dans toute l'Europe. D'autres pays ont apporté des réponses plus audacieuse en Espagne par exemple la loi. Entré en vigueur en août 2021 prévoit une présomption de salariat pour les livreurs à deux-roues et un droit d'accès des travailleurs à l'algorithme afin de conforter le mouvement juridisme jury se prudentielles en faveur de la requalification de certains travailleurs de plateforme. L'article 3 de la proposition de loi vise à introduire une distinction entre d'une part les véritables opérateur de mise en relation, et d'autre part les plateformes d'emploi qui exercent un contrôle juridique et économique sur les éléments essentiels de la relation au travail en conséquence travailleurs opérant en lien avec une plateforme devrait relever sous le contrôle du juge d'une relation de travail salarié et non du régime de la responsabilité sociale des plateformes en facilitant pour ceux qui le souhaitent la reconnaissance de leur lien de subordination avec les plateformes. Le texte a pour objectif de permettre à ces travailleurs de bénéficier d'une rémunération horaire minimal d'un encadrement des ruptures ainsi que d'une protection sociale Un mot du sort des travailleurs de plateforme sans papiers. Ceux-ci ont fait l'objet déconnection massive à la suite de la signature par les plateformes de livraison d'une charte relative à la lutte contre la forme la fraude et la sous-traitance irrégulière en outre ces travailleurs ne peuvent pas faute de bulletins de salaire à leur noms bénéficier des dispositions de la dit la circulaire du 29 novembre 2012. Dites circulaire Valls permettant la régularisation pour le travail, madame la ministre allez-vous permettent à ces travailleurs de sortir de l'impasse. a rejeté cette proposition de loi à titre personnel, je le regrette et espère que nos débats permettront de fédérer celles et ceux qui au sein de cette assemblée partage nos inquiétudes, je vous remercie. Merci cher collègue. La parole. Et maintenant Madame Carole Granjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Vous avez la parole madame la Ministre. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales Philippe mouiller. Monsieur le sénateur, Pascal Savoldelli madame la rapporteure Cathy ah pour se. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Nous ouvrons ce jour les débats sur la proposition de loi relative à la maîtrise de l'organisation algorithmique du travail de monsieur Pascal Savoldelli Madame Cathy ah pour polie et de leurs collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Je vous prie d'excuser l'absence du ministre du Travail Olivier Dussopt. Tout d'abord l'impact des algorithmes, sur l'organisation du travail est un enjeu important dont le gouvernement prend toute la mesure. Ce gouvernement et le ministre du Travail sont très attentifs aux mutations sociales entraînées par la révolution numérique. Nous avons lancé en décembre dernier. Les assises du travail visant à engager une réflexion sur le rapport au travail, la qualité de vie et la santé au travail, ainsi que la démocratie au travail. Ces assises ont réuni de manière large, les partenaires sociaux, des personnalités qualifiées et des universitaires. Ces travaux ont également inclus les questions liées au management par les algorithmes et des propositions seront formulées dans le rapport qui sera rendu dans les prochains jours. Par ailleurs, nous agissons également pour mieux réguler les relations entre les travailleurs des plateformes et les plateformes elles-mêmes ces dernières années un cadre juridique a été mis en place pour permettre l'émergence du dialogue social dans le secteur des plateformes de VTC et de livraison pour leur permettre de négocier un socle de droits ainsi nous saluons et je le salue en tant qu'ancienne un rapporteur sur le texte législatif. L'accord instaurant un revenu minimal de la course pour le secteur des VTC, qui témoigne de la dynamique engagée pour l'amélioration des droits sociaux des travailleurs de ce secteur d'activité. Bien sûr. Face aux métamorphoses du travail qu'implique la révolution numérique. Il faut accompagner et adapter notre modèle. Ainsi cette proposition de loi pose une question importante. Celle de notre rapport aux avancées technologiques. Il est donc important de rappeler que les contenus de ces technologies ne non pas de direction naturelle. Rien ne les destinant soit à contraindre le travail plutôt qu'à l'améliorer. Il nous revient de leur donner une intention de choisir comment mettre cette technologie à notre service. Disons-le clairement notre optimisme vis-à-vis de ces technologies n'est pas contradictoire avec une vigilance sur la forme des progrès qu'elle permet. À cet égard et contrairement à ce que certains voudraient faire croire, nous sommes attentifs à ce que l'homme continue de réguler et d'encadrer le travail pour ne pas céder à une administration ou une gouvernance par le les nombreux.

pour une meilleure organisation du travail. Je tiens à exprimer que nous ne pensons pas que cette proposition de loi donne une réponse satisfaisante à cette question. En effet, cette proposition de loi en proposant d'adapter les règles du droit du travail pour permettre. Pour mieux prendre en compte la gestion algorithmique pose en question en réalité d'une question. Qui met. Plus de difficultés. Sur la table qu'elle n'en résout. À cet égard, le gouvernement n'est pas la seule à le penser parce que mercredi dernier, la commission des affaires sociales du Sénat a rejeté cette proposition de loi. Ainsi la Commission partagent notre diagnostic sur l'utilité des dispositifs proposés revenons rapidement sur ces dispositifs présentés dans 3 articles d'abord le premier article propose de considérer les décisions ayant un effet sur les salariés et prise par un algorithme comme relevant de l'exercice du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur dans l'idée de le responsabiliser davantage face à une décision qui, qui l'aurait en réalité délégué un algorithme. Cette proposition n'ajoute en réalité rien à l'existant. De fait, la responsabilité de l'employeur n'est en aucun cas écartées par une prise de décision automatisée algorithmique. Pour le dire autrement un ordre passé par algorithme n'en est pas moins un indice de subordination à à l'employeur qui pourra être pris en compte par le juge pour prononcer une éventuelle requalification de la relation de travail. Il en va de même de l'autre proposition faite dans ce premier article de garantir l'accès du salarié aux décisions qui le concernent en matière disciplinaire et à leurs motivations dans l'idée d'instaurer une voie de recours humaine aux sanctions automatisé. De fait, le code du travail encadre déjà les procédures disciplinaires des entreprises et probablement mieux que ne le permettrait cette proposition plus précisément. Il n'est en droit du travail. Pas possible d'appliquer une sanction disciplinaire de manière automatique par un algorithme, d'autre part les voies de recours qui ne sont pas conditionner. Les voies de recours ne sont pas conditionnées au fondement de de la décision. Ainsi, si une sanction est prise sur le fondement de données récoltées par un algorithme. Les voies de recours ne sont pas différentes d'une décision prise sur la base d'informations purement humaine. Pour ne donner qu'un exemple. Face à une sanction le salarié peut systématiquement saisir le conseil de prud'hommes qui peut ensuite annulé la sanction si elle n'est pas justifiée à cet égard la proposition risque donc de rendre plus confus. Le droit existant plutôt que de l'améliorer. Ensuite le 2ème article propose qu'en cas de litige relatif à une discrimination indirecte les modalités de preuves soit aménagés il reviendrait ainsi à l'employeur d'apporter la preuve de l'absence de discrimination. Le motif est bien sûr louable. Nous savons que les algorithmes par définition aveugle à tout autre principe que l'optimisation sous contraintes peuvent entretenir des billets discriminant. Mais là encore je ne saurais dire à quel besoin. besoin. Cette proposition répond puisque le code du travail est unanime. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte sur la base de certains critères et ce peu importe le fondement de la discrimination et les moyens par laquelle cette discrimination ce produit. La charge de la preuve et déjà aménagé au bénéfice du salarié dès lors qu'elle allègue. D'une discrimination, y compris si cette discrimination et le résultat de l'utilisation d'un algorithme. Enfin le dernier article pose propose d'introduire dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de requalification de la relation entre un travailleur et une plateforme en écartant la qualification de plateforme de mise en relation. Dès lors que celle-ci exerce un contrôle juridique et économique sur les éléments essentiels de la relation de travail notamment par les moyens technologiques ou traitement automatisé là encore. Vous indiquez souhaiter inscrire dans la loi, le cadre jurisprudentiel existant de longue date sur la définition du lien de subordination. Cependant, la Cour de cassation n'a jamais retenu que l'exercice d'un contrôle juridique et économique y compris par des moyens technologiques ou traitement automatisé permettez de caractériser une relation de travail. À nouveau la solution proposée ne répond pas à l'ambition affichée, elle viendrait remettre en cause l'équilibre jurisprudentielle sur l'appréciation des critères de subordination, elle ne prend également pas en compte le cadre juridique défini depuis plusieurs années pour créer une véritable responsabilité sociale des plateformes et dont les acteurs se sont déjà emparés. En conclusion, comme je l'ai dit si nous partageons l'esprit de cette proposition de loi nous Noonan reconnaissons pas l'utilité et ne pouvons-nous le considérer comme une solution au management algorithmique. La priorité n'est donc pas de se précipiter sur l'encadrement des algorithmes, au risque de le faire maladroitement voire. Contre les protections déjà offertes par le code du travail dont l'application protège les travailleurs, il s'agit de redoubler de vigilance pour la bonne application du droit et de réfléchir plus avant à ce que l'on attend des algorithmes au travail je vous remercie. Merci madame la ministre je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 14h 50 pour la suite de l'examen de ce texte la séance. Suspendu.